J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la mission d'information sur Alstom et la stratégie industrielle du pays a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

d'abord, les deux chambres sont en désaccord sur les équilibres de finances publiques eux-mêmes. Le Sénat a adopté une trajectoire que nous jugeons moins ambitieuse, avec un ajustement structurel de 0,6 point en 2018, soit 12 milliards d'euros d'efforts supplémentaires à réaliser. Je dois à la vérité de vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement considère que ces chiffres ont peut-être été appréciés de manière rapide. En effet, que signifie un effort structurel fixé à 0,6 point de PIB pour nos concitoyens ? Cela signifie renoncer au dégrèvement de la taxe d'habitation ;

il resterait encore environ 5 milliards d'euros à documenter. Il s'agit donc, nous le voyons bien, d'une position qui relève plus de l'affirmation d'un positionnement politique que de la bonne gouvernance de nos finances publiques. Nous ne saurions y souscrire. À l'inverse, la majorité présidentielle, à l'Assemblée nationale, a voulu préserver les grands équilibres de ce texte et tenir ses engagements de campagne. Elle les finance et les rend effectifs, tout en maintenant le niveau d'ajustement structurel programmé en 2018 et les années suivantes. Je voulais aussi revenir sur la spécificité de nos discussions s'agissant des modalités d'association des collectivités territoriales au redressement des finances publiques. En effet, après les ajouts et les précisions de l'Assemblée nationale et du Sénat en première lecture, les propositions de la mission conduite par votre collègue Alain Richard et le préfet doivent permettre d'aller plus loin dans la définition du mécanisme de contractualisation et de reprise financière, dans le cadre de la concertation avec les élus et leurs représentants, concertation offerte et permise par la Conférence nationale des territoires. Certains d'entre vous étaient d'ailleurs présents à la Conférence nationale des territoires, qui s'est tenue à Cahors, jeudi dernier, sous la présidence du Premier ministre. Nous avons alors pu finaliser dans le dialogue la rédaction de l'amendement à l'article 10 dans la loi de programmation des finances publiques, telle que présentée aujourd'hui.

Je prendrai plusieurs exemples. La majorité sénatoriale a ainsi préféré hausser le plafond du quotient familial de 1 527 euros à 1 750 euros par demi-part pour l'impôt sur le revenu 2018, plutôt que de mettre en oeuvre, comme nous le proposons, le dégrèvement de la taxe d'habitation dès 2018. C'est un choix qui nous paraît d'autant plus surprenant qu'il repose sur le double constat, que nous partageons, de l'obsolescence de ses bases, ... Certes ! ... ainsi que de la nécessité de refonder, à terme, la fiscalité locale. La majorité sénatoriale a également fait le choix de supprimer la trajectoire carbone au-delà de 2018, tandis que l'Assemblée nationale l'a votée, consciente de l'urgence écologique à laquelle nous devons collectivement faire face. Là encore, c'est un choix politique. politique. Le Sénat a intégralement supprimé l'ISF, sans tenir compte de l'impact d'une suppression sèche de cet impôt, aussi bien sur les finances publiques que sur la structure elle-même de notre économie. Pour le dire autrement, l'idée d'une taxation différentielle de la rente au bénéfice de l'économie productive n'a pas recueilli votre assentiment, en dépit des atouts manifestes qu'elle nous semble présenter. Enfin, le Sénat a souhaité maintenir le niveau des crédits alloués aux collectivités territoriales dans le cadre de l'ancienne réserve parlementaire, tandis que l'Assemblée nationale avait explicitement prévu sa suppression. Au final, à l'issue de l'examen de la première partie, le solde budgétaire de l'État s'établissait à moins 86,4 milliards d'euros, soit une dégradation de 3,3 milliards d'euros par rapport à l'équilibre budgétaire présenté dans le projet de loi de finances, lequel tient compte, il est vrai, de l'impact de l'annulation de la taxe à 3 % sur les dividendes. Troisième cause de l'échec des CMP, et non des moindres : l'examen de la seconde partie de projet de loi de finances. Comme vous le savez, l'ensemble des votes intervenus sur la seconde partie du projet de loi de finances a conduit, à la suite notamment du rejet des crédits de cinq missions du budget général,

Sur la mission « Travail et emploi », je tiens en particulier à rappeler que le Gouvernement triple l'effort budgétaire en faveur de la formation des jeunes et des chômeurs de longue durée. Sur la mission « Sécurités », nous regrettons l'attitude qui consiste à la fois à reprocher au Gouvernement une hausse insuffisante des crédits de la mission et à décider de n'en voter aucun. Concernant Concernant la mission « Justice », le budget proposé est en hausse de quasiment 4 %, comprenant notamment une augmentation de presque 5 % des crédits de fonctionnement, d'investissement et d'intervention, et la création d'un millier d'emplois.

Je tiens d'ailleurs à rappeler l'événement important qui s'est produit jeudi dernier dans ce dossier : la signature, entre le Gouvernement et une partie substantielle du mouvement HLM- représentant plus de 40 % du parc locatif social -, d'un protocole d'accord sur la base du texte que nous vous présentons aujourd'hui. Pour conclure, j'aimerais évoquer avec vous une série de convergences qui méritent, malgré tout, d'être relevées. Je pense tout d'abord à l'avenir de la réforme de la procédure parlementaire conduisant au vote de la loi de finances, notamment au rapprochement de la discussion des dispositions relatives aux recettes, qu'elles soient fiscales ou sociales, lequel, selon le rapporteur général pourrait permettre au Parlement de porter un regard plus éclairé sur la cohérence d'ensemble de la politique du Gouvernement en matière de prélèvements obligatoires ». Au-delà de cette remarque procédurale, il suffit de parcourir les différents rapports sénatoriaux sur ces deux textes pour se convaincre des points d'accord qui existent entre les deux chambres. Là encore, je prendrai plusieurs exemples. Au sujet de la sincérité de ce projet de loi de finances, le rapporteur général indique, dans le tome I de son rapport, que « le Gouvernement semble s'engager à revenir à une pratique plus conforme au principe de l'autorisation parlementaire des dépenses Si l'on regarde les différentes missions du budget général, je note par ailleurs, à titre d'illustration, que, selon le rapporteur spécial de la mission « Défense », « le budget 2018 comporte différents motifs de satisfaction et devrait permettre de répondre globalement aux besoins des armées Emmanuel Capus, rapporteur spécial de la mission « Travail et emploi », les crédits de la mission « seront maintenus à un niveau très élevé » et « permettront le financement des dispositifs en faveur de l'emploi des jeunes et des personnes les moins qualifiées en particulier, la montée en puissance de la garantie jeunes et le lancement du plan d'investissement dans les compétences Au-delà, à propos des contrats aidés, dont la diminution du volume contribue certes au redressement de nos comptes publics mais peut nourrir des inquiétudes, le rapporteur spécial s'exprime en des termes que nous pourrions partager quand il indique que, « sans contester l'utilité de ces emplois pour les collectivités territoriales et le secteur associatif, ceux-ci ne constituent pas moins des contrats précaires subventionnés et, partant, une réponse de court terme, parfois motivée par des raisons purement statistiques Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, par-delà les positionnements de chacune des deux assemblées et les lignes de partage idéologiques, il y a des prises de position responsables qui, de part et d'autre, auraient pu laisser penser à l'aboutissement d'un consensus, fût-il ponctuel et parcellaire, avec la majorité sénatoriale.

2018 à 2022. Vous le savez, des divergences importantes sont apparues entre nos deux assemblées. Elles ont conduit, à notre grand regret, à l'échec des deux commissions mixtes paritaires, qui se sont déroulées le 13 décembre dernier.

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause la création de l'impôt sur la fortune immobilière, dont le périmètre est pour le moins incompréhensible, puisque les liquidités, les bitcoins ou les diamants, autant de placements

Je pense à la responsabilité solidaire des plateformes de commerce en ligne pour le paiement de la TVA. Je ne comprends pas cette position. Il s'agit en l'espèce d'une fraude avérée à la TVA. Nous nous étions inspirés d'un dispositif qui fonctionne au Royaume-Uni,

Ainsi, je me félicite de l'adoption de l'article 8 introduit sur notre initiative, qui rappelle les engagements du Président de la République en matière de réduction d'emplois de l'État et de ses opérateurs sur la période quadriennale. Je me félicite également de la reprise des dispositions

Le double discours permanent et le brouillage des repères sont une marque de fabrique qu'il convient de dénoncer. En outre, ce qui caractérise l'action du Gouvernement, c'est souvent la brutalité l'impréparation avec laquelle il conçoit les réformes structurelles. Comme si, pour faire bouger notre pays raillé pour son immobilisme, il fallait commencer par détruire violemment l'existant, sans avoir construit auparavant les bases d'une alternative crédible. Fait majeur, ce budget va approfondir les inégalités et affaiblir notre modèle social. Au nom d'un monde nouveau, il nous propose un vaste retour en arrière, à rebours de la décentralisation, engageant des réformes portant le sceau des politiques libérales mises en oeuvre dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix qui, on le sait de manière encore plus documentée depuis quelques jours, ont produit une augmentation massive des inégalités. Le « premier de cordée » monte toujours plus haut, équipé jusqu'au bout des doigts, assuré par son capital financier, social et culturel, mais il laisse en bas celui qu'il accuse de n'être pas assez combatif pour grimper, alors que ce dernier ne dispose que de la simple force de ses bras. Double discours, méthode brutale et augmentation des inégalités sont donc les caractéristiques de ce budget. L'ultra-communication permanente de ce gouvernement ne saurait nous faire oublier une certaine dualité dans le discours. Vous dites vouloir lutter, à l'échelon européen, contre l'évasion fiscale, monsieur le secrétaire d'État, mais vous ne saisissez pas nos propositions pour agir dès maintenant. Prenons l'exemple de la fraude à la TVA pour les plateformes ou de la taxation des GAFA. Pourquoi ne reprenez-vous pas ces propositions votées ici, au Sénat, et de façon consensuelle ? Vous prétendez lutter, à l'échelon européen, contre le fiscal, mais vous jouez le jeu du nivellement par le bas, en essayant d'atteindre une moyenne européenne que nos voisins s'empresseront bien vite de faire baisser à nouveau. Vous dites vouloir mettre en oeuvre un Grand plan d'investissement. Or il n'apparaît pas, ou peu, en crédits de paiement : moins de 2 milliards d'euros pour 2018, quand vous annoncez 57 milliards d'euros Vous vous targuez de présenter un budget responsable, mais ce budget cache en réalité un vaste plan social, relativement silencieux, que l'État mène dans ses administrations et ses agences. Je pense à l'INRS ; je pense à l'INSEE ; je pense à Pôle emploi je pense à l'AEFE ; je pense aussi à la DIRECCTE, à l'IRSTEA, à Météo France, à France Télévisions, et j'en passe. Au-delà du double discours, il y a aussi l'utilisation récurrente d'une méthode brutale qui consiste à casser un système avant même de préparer la construction du suivant.

plutôt que d'annoncer une grande réforme du logement et de faire passer des mesures budgétaires qui risquent de provoquer un effondrement de l'offre, vous aviez pris le temps de mettre en place une véritable concertation avec les bailleurs sociaux et avec

vous en supprimez une large part. Vous précarisez des personnes éloignées de l'emploi, pour qui la réinsertion professionnelle, et donc sociale, était concrète. Vous déstabilisez les collectivités territoriales et les associations dans la mise en oeuvre de leurs actions. En contrepoint, vous annoncez une grande réforme de la formation professionnelle,

Vous souhaitez aussi contrôler leurs dépenses, à travers la contractualisation que les préfets vont mettre en oeuvre, rétablissant de ce fait le contrôle des budgets des collectivités.

même brutalité a aussi obligé le Premier ministre à faire des modifications importantes sur la contractualisation, allant bien au-delà de la simple précision. N'aurait-il pas été plus raisonnable de commencer par là ? Une réflexion large et collective aurait certainement permis d'éviter l'arrivée dans le débat parlementaire, au stade de la nouvelle lecture, du nouveau dispositif de contractualisation liant l'État et les collectivités. S'agissant d'une mesure aussi importante, est-il acceptable que le travail parlementaire soit ainsi réduit à une heure pour l'Assemblée nationale et une journée pour le Sénat ? Je veux m'arrêter ici quelques instants sur les modifications introduites dans le projet de loi de programmation des finances Sur le fond de l'article 24, l'exclusion d'une partie des dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité peut apparaître à première vue comme une avancée pour les départements. Mais ici on retrouve le double discours, car, en réalité, l'objectif de réduction, la cible finale de 13 milliards d'euros, est maintenu Si ces dépenses ne sont pas intégrées dans l'effort à fournir, celui-ci devra donc être concédé sur d'autres postes de dépenses départementales, ou reporté sur d'autres collectivités le mécanisme de correction, auparavant uniquement mentionné dans son principe, il est maintenant précisé. Au final, votre démarche est habile, mais ne nous leurrons pas sur son résultat. L'objectif de contenir les dépenses de fonctionnement à 1,2 en valeur, c'est-à-dire au niveau de l'inflation les premières années et en deçà du niveau de l'inflation en fin de période de programmation, ne pourra que conduire à des efforts de réduction des dépenses considérables pour les collectivités territoriales. Cela ne manquera pas d'affaiblir le service public local. Aux mesures impréparées, sinon brutales, s'ajoutent des mesures fiscales injustes, qui entraîneront inexorablement un accroissement des inégalités. Après avoir augmenté la CSG, vous décidez de supprimer la presque totalité de l'impôt de solidarité sur la fortune, et de mettre en place une pour les revenus du capital ; je note d'ailleurs que l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement du Sénat visant à éviter l'optimisation fiscale qui en découlera et qui risque de coûter beaucoup plus cher

Accroissement des inégalités, toujours : qui va payer l'augmentation de la fiscalité écologique ? Ce sont les bas revenus qui dépassent le seuil très bas de l'accès au chèque énergie, soit 7 700 euros par an et par unité de consommation. Les effets positifs d'une fiscalité écologique seront socialement injustes. Ainsi, vous réduisez la part des efforts demandés aux plus riches, vous accentuez celle demandée aux plus modestes et, dans le même temps, vous affaiblissez les services publics. La pression que vous mettez sur les collectivités et certains ministères va fragiliser les services publics essentiels. Les réduire va inexorablement conduire à une augmentation des inégalités. Nous ne pouvons pas agir comme si nous ignorions que la baisse de la fiscalité des hauts revenus s'accompagnait toujours d'un accroissement des inégalités. Le dernier rapport des économistes autour de Thomas Piketty nous le confirme. Que de références ! Sur le long terme, l'économie ne peut bien fonctionner que si la croissance est équitablement répartie. Le modèle français repose sur une redistribution des revenus après impôt et sur un accès à la protection sociale et aux services publics. En copiant le modèle anglo-saxon- fiscalité favorable aux plus riches, flexibilisation du marché du travail, etc. -, vous attaquez l'équilibre de notre système. Pour quelques hypothétiques points de PIB, vous orientez notre société vers plus de précarité et d'inégalités. Mes chers collègues, face à ce budget initialement marqué à droite, la majorité sénatoriale a pratiqué

Le risque, ce n'est qu'un jeu pour ceux qui ont un patrimoine bien garni, un carnet d'adresses bien rempli, des diplômes bien fournis. Mais le risque peut aussi être un voyage sans retour vers la pauvreté pour ceux qui n'ont comme filet de sécurité que la sécurité sociale et comme unique patrimoine le service public.

les projets de loi de programmation des finances publiques pour la période 2018-2022 et de loi de finances pour 2018. À nouveau, et malheureusement sans surprise, les deux commissions mixtes paritaires n'ont pu se mettre d'accord sur les articles restant en discussion. Ce blocage nous laisse un goût d'occasion manquée. Dans le cas du projet de loi de finances, nous avions déploré que le Sénat adopte une position de principe et renonce à l'opportunité d'améliorer le texte dans un sens acceptable par la majorité présidentielle. Nous regrettons également que l'Assemblée nationale ait supprimé de bonnes mesures, adoptées par notre assemblée sous les auspices du rapporteur général, telles que le rehaussement du plafond du quotient familial ou les dispositions concernant la fiscalité du numérique. Nous saluons toutefois l'adoption définitive de certains des amendements que nous avions déposés : ceux relatifs à la fiscalité énergétique ; l'amendement sur les critères de classement en zone de revitalisation rurale, cher à notre collègue Alain Marc ; l'amendement sur l'assurance des installations d'énergie marine renouvelable. Notre groupe a ainsi pleinement contribué à l'élaboration de ce projet de loi de finances. Nous espérions que cette seconde lecture puisse sauver ce qui pouvait encore l'être et qu'elle soit l'occasion d'un débat plus apaisé. Il semble que tel ne sera pas le cas. Je ne reviendrai pas sur le projet de loi de finances pour 2018. Il a déjà fait l'objet de nombreux débats et nous a permis d'exposer maintes fois notre position en faveur d'une approche constructive, équilibrée et pragmatique des différentes réformes envisagées. Nous avons toujours la même exigence aujourd'hui : l'équilibre entre la création de l'IFI, l'instauration de la et le dégrèvement de la taxe d'habitation est certes imparfait, mais il constitue un compromis politique et économique robuste entre la nécessité de réorienter l'épargne vers notre économie et la restitution de pouvoir d'achat à nos concitoyens. C'est également un équilibre fragile. Le Sénat l'a déjà rompu au détriment des classes populaires et des classes moyennes. Nous n'aurions pu que nous opposer à une nouvelle tentative allant dans ce sens. La nouvelle version du projet de loi de programmation des finances publiques contient, elle, des nouveautés substantielles. La Conférence nationale des territoires, enceinte nouvelle qui semble permettre de vraies avancées de fond, a débouché sur deux amendements du Gouvernement. Si on peut déplorer le caractère précipité et tardif de leur dépôt, ils traduisent néanmoins des discussions de longue haleine qui ont eu lieu ici même au Sénat, à l'Assemblée nationale, entre les associations d'élus et le Gouvernement, et dans le cadre, enfin, de la mission conduite par notre collègue Alain Richard et Dominique Bur. C'est l'honneur du Premier ministre, Édouard Philippe, que d'avoir su écouter et entendre les différentes parties prenantes pour proposer un mécanisme de contractualisation plus respectueux des réalités locales et des propositions faites par notre assemblée. Je note que M. le rapporteur général vient d'indiquer que des portes avaient été entrouvertes ; c'est tout dire ! Nous pensons que plusieurs décisions vont dans le bon sens. Par exemple, les nouvelles marges de souplesse autour du taux d'évolution standard des dépenses de fonctionnement constituent incontestablement un instrument de flexibilité bienvenu. Le « bonus » accordé aux collectivités respectant les objectifs fixés, sous forme de bonification des dotations d'investissement, constitue une incitation à la vertu et rompt avec la logique essentiellement punitive du précédent texte. L'abandon de la « règle d'or renforcée » contenue dans la première version du projet de loi de programmation, qui prévoyait le déclenchement d'une procédure de surveillance des collectivités dont le rapport entre l'encours de dette et l'épargne brute dépassait les onze à treize ans, est quant à elle une mesure de bon sens, plus favorable à l'investissement. La meilleure prise en compte, enfin, de la structure des dépenses des départements pour tenir compte de leur dynamique particulière semble constituer une reconnaissance opportune des spécificités propres aux différents niveaux de collectivités. Tous ces éléments sont le fruit d'une méthode de gouvernement qui nous convient : concertation, analyse et action résolue. Néanmoins, nous croyons que la logique consistant à faire peser lourdement l'effort de maîtrise de la dépense publique sur les collectivités locales manque son but. D'une part, elle méconnaît la dynamique de la dépense et de l'endettement, qui est d'autant plus problématique au niveau de l'État et des organismes de sécurité sociale. D'autre part, elle masque le fait que les efforts inscrits dans cette loi de programmation sont globalement insuffisants pour combler notre retard sur les autres pays de la zone euro, et en particulier sur l'Allemagne. Cela ne signifie pas que les collectivités doivent être exemptées de l'effort national d'assainissement des finances publiques. Elles doivent prendre leur juste part, et elles en ont conscience. Cela signifie qu'il ne faut pas se tromper de combat et que d'autres priorités devraient figurer, monsieur le secrétaire d'État, en haut de votre agenda. Je veux parler de la baisse des effectifs dans la fonction publique, de l'effort de l'effort structurel en dépense, trop faible pour réduire durablement le déficit public, et, enfin, du désendettement de l'État, qui devrait, lui, faire l'objet des fameuses « règles d'or renforcées Ces deux textes constituent donc un premier pas en direction du nouveau monde de sincérité et de responsabilité qu'on nous a promis. Néanmoins, ils prouvent également que ce nouveau monde ne se décrète pas : il se construira patiemment, résolument, à force de courage et dans l'action.

par certaines des dispositions qui ont été votées. Je le répète, l'augmentation de 40 % des indemnités des maires de grande ville et des présidents de conseil départemental ne passe absolument pas

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, autant le dire d'emblée : je regrette que les commissions mixtes paritaires ne soient pas parvenues à établir des versions communes du projet de loi de finances et du projet de loi de programmation.

L'absence d'accord avec l'Assemblée nationale empêchera, malheureusement, qu'une grande partie de ce travail trouve une juste concrétisation. Vendredi, les députés ont rétabli leurs versions des projets de loi et supprimé la plupart des modifications apportées par la Haute Assemblée, notamment celles adoptées sur l'initiative de mon groupe.

ont dès le début fait consensus, comme la réduction du taux d'impôt sur les sociétés, aucun accord n'a été trouvé sur les mesures les plus emblématiques, qui sont aussi celles auxquelles nos concitoyens sont particulièrement sensibles dégrèvement de la taxe d'habitation,, impôt sur la fortune immobilière, contractualisation, etc. Sur des sujets moins médiatiques, comme la compensation de la taxe professionnelle, les agences de l'eau ou les réseaux consulaires, il n'y a pas eu davantage d'accords.

au coeur de la puissance publique -, elle s'est elle-même privée de proposer un véritable budget alternatif et responsable. Je le regrette très profondément. Pour ce qui concerne les grandeurs macroéconomiques, le déficit public s'établirait l'an prochain à 2,8 % du PIB, contre 2,9 % attendus cette année. La trajectoire à l'horizon 2022 prévoit une poursuite de la baisse, concentrée toutefois sur la fin du quinquennat, avec une remontée en 2019, du fait de latransformation du crédit d'impôt pour Cette évolution globalement positive, quoique modeste dans son ambition, reste tributaire des évolutions de la conjoncture et de chocs contentieux, comme l'invalidation de la taxe additionnelle sur les dividendes. Les réformes de la taxe d'habitation et de l'impôt sur la fortune auront concentré l'attention des médias. Le dégrèvement de la taxe d'habitation continue de susciter une vive opposition

En outre, la réforme ne résout pas vraiment le problème des bases, qui servent toujours au calcul des taxes foncières. À quand une vraie remise à plat du système fiscal local ? Enfin, la question des compensations reste en suspens. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, remplacé par la seule imposition du patrimoine immobilier, est l'une des mesures les plus clivantes du texte. Son coût n'est pas négligeable, puisqu'il s'élèverait à quelque 4 milliards d'euros dès l'an prochain. La transformation de l'ISF en IFI doit créer un choc d'attractivité. Il est vrai que si les paradis fiscaux ont fait beaucoup parler d'eux dernièrement, à juste titre, la France véhicule aussi- il faut le reconnaître -l'image d'un pays tributaire d'un système fiscal lourd et complexe. Le radical de coeur que je suis, attaché à la dimension citoyenne de l'impôt, ne peut que se désoler de cette situation. Toutefois, le Gouvernement devrait être plus soucieux de stabilité fiscale. Concernant la programmation pour 2018-2022, les principales mesures, à savoir les articles 10 et 24, sont toujours en discussion. En première lecture, le Sénat avait pourtant apporté des précisions utiles au principe de contractualisation. Il avait notamment donné des garanties aux collectivités en imposant des engagements financiers de la part de l'État. La règle d'or « renforcée » avait été supprimée, car jugée injustifiée alors que l'endettement des collectivités territoriales ne représente qu'une faible partie de l'endettement public. Ce matin, la commission des finances, dans son immense sagesse, a partiellement rétabli son texte de première lecture. Nous réexaminerons tout à l'heure ce projet de loi, auquel le RDSE est favorable, en espérant trouver davantage de points d'accord avec l'Assemblée nationale. Néanmoins, je veux saluer les aspects indéniablement positifs du projet de loi de finances, tels que le maintien et même la légère augmentation des dotations aux collectivités, qui contrastent avec l'austérité du quinquennat précédent, les progrès introduits dans l'imposition des plateformes internet et des entreprises du numérique, mais aussi la poursuite du soutien à l'investissement public local ... Sur le projet de loi finances, la commission a choisi de présenter une motion tendant à opposer la question préalable. Le RDSE est opposé par principe à ce dispositif

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, il est trop tard dans la procédure parlementaire pour « refaire le match » sur ces deux textes complémentaires : le projet de loi de finances pour 2018 et la trajectoire pluriannuelle des finances publiques 2018-2022. Leurs commissions mixtes paritaires respectives ont échoué, et nous revoilà en nouvelle lecture où rien ne se dira, je le crains, de bien neuf, car les positions sont à présent claires. Tout d'abord, la majorité sénatoriale a décidé de voter un projet de loi de finances à la découpe. La fiscalité du capital ? On prend. La réforme de la taxe d'habitation ? On ne prend pas. La fiscalité des entreprises et la transformation du CICE ? On prend. Le budget de la mission « Travail et emploi » et les crédits en faveur de l'apprentissage ? On ne prend pas. Cela clignote comme une guirlande de Noël, maiscela sent surtout le sapin pour notre débat qui risque hélas ! d'être victime

affichée de réduire davantage les déficits et la crédibilité des pistes d'économies du côté de la majorité sénatoriale. Par piste d'économies, je n'entends pas les milliards d'euros de réduction du fait du rejet de cinq budgets, mais des propositions de maîtrise plus solides et surtout plus plausibles. Nous n'approuvons pas cette politique du rabot qui n'a pas fait ses preuves dans le passé, qui a d'ailleurs été une des limites de la révision générale des politiques publiques et qui, je le crois, peut même nourrir la défiance de nos concitoyens- au même titre que l'excès de dépense publique est de nature, elle aussi, à faire naître le scepticisme, car la qualité de certains services publics n'est pas à la hauteur des attentes, et ce non par absence de ressources, mais parce que leur gestion pourrait être plus efficace. La confiance ne se décrète pas, mes chers collègues, mais elle peut néanmoins être encouragée par certains choix politiques. La Conférence nationale des territoires, qui s'est tenue jeudi dernier à Cahors, en est une illustration. Elle mérite que l'on s'y attarde un peu, en particulier au sein de notre assemblée, parce que ses conclusions ont modifié l'autre texte, celui relatif à la trajectoire des finances publiques. Les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales ont besoin d'être rénovées. Encore une fois, il aurait été plus facile d'annoncer une baisse aride et injuste des dotations pour 2018, 2019 et 2020. Une partie de notre assemblée fait mine d'avoir oublié la période dont nous sortons à peine. Le Gouvernement a préféré dialoguer et contractualiser la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour les 340 collectivités dont le budget excède 60 millions d'euros. Qu'il me soit permis ici de saluer le remarquable travail mené par notre collègue Alain Richard et le préfet Dominique Bur à la demande du Premier ministre, dans un délai contraint et sur un sujet aussi délicat. Concrètement, 99 % des collectivités ne sont pas concernées par cette contractualisation. Plutôt que de pousser avec retard des cris d'orfraie, alors que les coupes aveugles dans les dotations se sont arrêtées, soyons collectivement au rendez-vous de ce nouveau pacte financier. La contractualisation qui devra intervenir au premier semestre 2018 reposera sur un objectif contraignant de maîtrise des dépenses de fonctionnement- les fameux 1,2 % refusés ici -, objectif qui pourra être adapté en fonction de la situation de la collectivité et sur deux objectifs indicatifs, à savoir l'évolution du besoin de financement et la trajectoire de désendettement. La confiance n'exclut pas le contrôle : cela ne me choque pas qu'une collectivité ne respectant pas sa trajectoire de maîtrise de dépenses se voie opposer un mécanisme de correction. Très concrètement, la collectivité se verrait appliquer une reprise financière de 75 % du dépassement, dans la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement. Il faut noter que pour les collectivités refusant d'entrée de jeu de contractualiser avec l'État, la reprise financière s'élèverait à 100 % du dépassement, ce qui constitue une incitation persuasive. Que l'on puisse critiquer tel ou tel aspect du dispositif retenu, je le conçois, c'est le jeu. Mais on ne peut pas mégoter ou chipoter chaque fois qu'une proposition est sur la table, sauf à tenir un double discours qui consiste, en réalité, à s'opposer à toute forme encadrée de maîtrise de la dépense locale. Le dialogue continue, il porte et portera encore ses fruits. Par exemple, les préoccupations des départements en matière d'allocations individuelles de solidarité ont été entendues par le Gouvernement, et c'est pourquoi une partie des dépenses de solidarité seront exclues de l'objectif de 1,2 % d'évolution Dominique Bussereau, qui n'est pas éloigné de la majorité sénatoriale, a salué cette évolution. L'État a bien conscience que la situation financière de certains départements doit être assainie. C'est pourquoi le collectif budgétaire prévoit un fonds exceptionnel de 100 millions d'euros. L'Assemblée des communautés de France, présidée par Jean-Luc Rigaut, lui aussi peu éloigné de vos travées, a appelé ses membres à contractualiser avec l'État. Pour les régions, Hervé Morin est revenu à la table des négociations et a estimé qu'il y avait désormais une base de discussion acceptable entre l'État et les régions. Jean-Luc Moudenc, qui me semble avoir l'étiquette Les Républicains et qui préside France Urbaine, s'est montré favorable aux annonces de Cahors. Alors oui, une partie de l'Association des maires de France est déjà en campagne municipale, en tout cas certains de ses dirigeants historiques. D'autres sont plus constructifs, comme en atteste la mission sur l'évolution de la fonction publique territoriale que vous aviez confiée, monsieur le secrétaire d'État, à Philippe Laurent. Le Premier ministre n'a pas parlé que de froideur comptable dans le hangar glacial de Cahors, mais aussi de projets ambitieux un nouvel élan pour améliorer l'accès à internet pour nos territoires ruraux, un assouplissement du calendrier de transfert de la compétence eau, un plan de 5 milliards d'euros pour revitaliser le centre des villes moyennes, ou encore l'encouragement à l'expérimentation au niveau local. Ces textes rendent possible une vraie décentralisation, que nous appelons de nos voeux. Reconnaissons que nous avons plutôt assisté au cours de la dernière décennie à un long entracte. La République a rendez-vous avec ses territoires, comme nous le verrons en 2018. Ce projet en pose les premières

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la loi de finances pour 2018 porte clairement la signature de la nouvelle majorité présidentielle. Mais, plus que tout, elle n'est que la première « levée » de la loi de programmation.

Le premier élément, c'est le carcan de l'Union européenne : tant dans la loi de programmation que dans la loi de finances, il faut se conformer aux règles fixées par la Commission européenne. même Commission qui a fait du rêve européen le cauchemar d'une société inégalitaire, d'une croissance aux fruits mal partagés, d'une puissance centrifuge qui pèse sur la souveraineté de notre peuple comme sur l'unité de certains de pays membres. L'Europe ne sait même pas lutter contre la fraude fiscale qui se déroule sous ses yeux, et même dans son arrière-cour. Cette Europe, qui n'est toujours pas sociale, est suspendue au fil de la finance. Venons-en au deuxième élément, celui qui, telle la deuxième mâchoire de l'étau, unit les deux textes : l'appétit des marchés financiers. Parce que c'est bien beau les critères européens, la convergence des politiques publiques et budgétaires, etc. Mais il faut tout de même dégager des marges pour que les marchés y trouvent leur compte ... Et force est de constater que le tribut électoral exigé par les marchés financiers qui ont fait élire Emmanuel Macron a été largement payé. Il y a, d'abord, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune : ce cadeau de 5 milliards d'euros aux plus riches coûtera 15 000 euros par contribuable concerné ! Il y a, ensuite, le prélèvement forfaitaire unique. Nous n'avons pas vraiment goûté cette disposition, qui nous a semblé offrir aux revenus du capital un avantage fiscal inconsidéré. Ce prélèvement, c'est un peu ! Rappelez-vous,

Ce PFU, que vous avez approuvé, m'a paru bien plus fort que l'ISF-PME de Nicolas Sarkozy ou son relèvement des plafonds d'exonération des donations, et bien plus fort encore qu'Édouard Balladur et ses stock-options sans délai de portage minimal. minimal. Mes chers collègues, la grande nouveauté du PFU, c'est de reproduire le schéma exact de l'avoir fiscal de Valéry Giscard d'Estaing, issu de la loi du 12 juillet 1965 ... Quelle innovation

faciliter le développement de l'épargne et le financement des investissements ; permettre de reconstituer un marché financier contribuant activement à l'équipement du pays ; faire disparaître les obstacles qui contrarient le développement et la rénovation des structures industrielles. » industrielles. » Monsieur Bargeton, toute ressemblance du discours d'hier avec celui d'aujourd'hui n'est sans doute que pure coïncidence ! Monsieur le rapporteur général, par un amendement dont je ne suis pas certain qu'il sera retenu par l'Assemblée nationale, vous avez voulu mettre en place un système anti-abus, pour éviter que l'incitation à se payer en actions ne soit trop forte. Vous avez notamment visé les cadres dirigeants d'entreprise et vous êtes interrogé sur leur taux de détention du capital. Vous avez fixé de fait une norme à 10 % de ce dernier.

même si Franck Riboud aura touché en 2016 plus de 540 000 euros de dividendes, s'ajoutant aux 2 petits millions d'euros de sa rémunération fixe annuelle ... Paradoxalement, monsieur le rapporteur général, ce sont plutôt les PDG de grosses PME ou d'entreprises de taille intermédiaire qui seraient gênés aux entournures par les mesures que vous préconisez.

Elle aura donc été entendue par le nouveau Président de la République et son « nouveau monde », un président dont les promesses semblent ainsi venir de quelques rangs poussiéreux. La nouveauté tarde à se manifester ! La discussion de la seconde partie du budget n'a pas été meilleure. J'en garde un souvenir particulier

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous partageons pour l'essentiel les grands objectifs de ce budget sous-tendu par la force de la volonté politique et des engagements tenus : maîtrise de la dépense publique, résorption des déficits, désendettement du pays, orientation de l'épargne vers le financement de nos entreprises en vue d'ouvrir une nouvelle voie pour tenter de relever le défi de l'emploi quand tant d'autres solutions ont montré leurs limites, stabilisation des concours financiers aux collectivités territoriales. En première lecture, le Sénat a conduit un travail de fond, apportant des améliorations qui nous semblaient justes, aux uns et aux autres, en fonction de nos sensibilités et de la connaissance que chacun d'entre nous a des réalités du terrain. Cela a été dit, de nombreux articles ont pu être votés conformes par les deux assemblées. Toutefois, le débat a aussi mis en évidence des divergences sur des points essentiels qui ont rassemblé une majorité de sénateurs et rendent aujourd'hui un accord global impossible. Pour ma part, je regrette- je le dis en toute objectivité -qu'un certain nombre de mesures adoptées par le Sénat, parfois simples

qui, vous le savez, me tient à coeur : le prêt à taux zéro, pour lequel nous demandions un traitement équitable de tous les primo-accédants, qu'ils soient ruraux ou urbains

D'une façon plus générale, monsieur le secrétaire d'État, le groupe Union Centriste est attaché à des valeurs sur lesquelles nous ne transigerons pas, mais sur le fondement desquelles nous pourrons aussi vous apporter un soutien sans équivoque.

C'est même une des missions essentielles de l'État que de veiller à ce que les transformations de notre société ne laissent pas au bord du chemin les moins agiles ou les plus fragiles de nos concitoyens.

Je crois pouvoir dire que nous partageons cette analyse, mais nous divergeons manifestement non seulement sur l'intensité et la profondeur de la rupture nécessaire, mais aussi sur les moyens L'examen de ce premier budget du quinquennat le démontre à l'évidence. Du fait de son manque d'ambition, celui-ci ne peut constituer l'amorce du redressement dont la France a besoin. Trois éléments suffisent à le démontrer en 2018, les dépenses de l'État continueront de progresser ; le déficit du budget également, de près de 7 milliards d'euros ; quant à la réduction du nombre de fonctionnaires, elle sera limitée à 1 600 dans le périmètre de l'État.

il nous faut relancer l'économie en créant un véritable choc de compétitivité par une baisse massive de charges de nature à redonner des marges à nos entreprises, sans lesquelles toute amélioration durable sur le front de l'emploi est hors D'autre part., il nous faut stabiliser, voire diminuer, les impôts et taxes pesant sur les ménages, notamment ceux qui ont été le plus touchés depuis 2012 par des hausses massives de la fiscalité. du sempiternel débat opposant politique de l'offre et politique de la demande, nous affirmons qu'il est urgent de mener les deux conjointement. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé des mesures en faveur de nos entreprises, des PME, de l'innovation, mais aussi du pouvoir d'achat des retraités, des familles et des propriétaires, notamment, grands oubliés de votre politique. Mais il nous faut aussi, et c'est bien là que les choses se compliquent, réduire fortement notre déficit public, afin d'enrayer la spirale infernale d'une dette qui ne cesse d'augmenter et nous menace toujours comme une épée de Damoclès.

Nous ne considérons pas que la dépense publique soit, par nature, toujours trop élevée, mais, à l'évidence, nous ne pouvons plus la financer par l'emprunt ou par l'impôt. Nous le savons, revenir à l'équilibre des comptes publics demandera des efforts importants. Cependant, l'Allemagne l'a fait : pourquoi en serions-nous incapables ? Malheureusement, l'effort est reporté en fin de quinquennat et les mesures annoncées sont toujours aussi faiblement documentées. C'est pourquoi nous avions proposé des mesures importantes d'économies dès l'an prochain. Or rien n'a été retenu par l'Assemblée nationale. Après une commission mixte paritaire écourtée, nous avons assisté à un détricotage en règle, par les députés de La République En Marche, de l'ensemble des mesures adoptées par le Sénat, qui a eu manifestement le grand tort de ne pas s'aligner sur la ligne imposée par l'exécutif. monde » dont l'émergence a été claironnée, à grand renfort de communication, où est cet esprit « constructif » quand la majorité présidentielle supprime méticuleusement toutes les mesures adoptées par l'autre chambre, y compris celles qui l'ont été à la quasi-unanimité ? Je pense par exemple aux mesures relatives à l'économie collaborative, qui est ici un sujet consensuel. Même notre article visant à lutter contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne a été supprimé, alors qu'il avait été adopté à l'unanimité, y compris donc par les sénateurs de La République En Marche, avec un avis de sagesse du Gouvernement ! C'est à n'y rien comprendre comprendre ! Nous avons bien compris que les députés de La République En Marche avaient très peu de marge de manoeuvre. Le Sénat est-il donc également considéré comme une simple chambre d'enregistrement ?

Le seul apport du Sénat aura donc été de transcrire le recours à une augmentation de la TVA à hauteur de 700 millions d'euros, ce que l'Assemblée nationale n'avait pas eu le temps de faire, puisque l'idée avait été avancée lors de l'examen en première lecture de la seconde partie du projet de

Et comment ne pas pointer le ridicule de la mesure qui a finalement été retenue par l'Assemblée nationale ? L'APL accession est en fait maintenue, pour deux ans seulement, mais en zone III, c'est-à-dire en zone détendue,

? Comment ne pas pointer l'incohérence de vos décisions en matière de logement ? Vous allez ponctionner, par la baisse des loyers, de 1,7 milliard à

De l'autre côté, vous incitez ces mêmes bailleurs à vendre 40 000 logements par an pour retrouver des fonds propres, puisque vous leur en retirez, et vous supprimez l'APL accession. Voilà une vraie politique de gribouille sur un sujet pourtant essentiel pour notre économie et pour les Français

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le projet de loi de programmation des finances publiques a été très substantiellement modifié en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, au lendemain de la Conférence nationale des territoires, qui s'est tenue le 14 décembre dernier. La contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales a été précisée. En première lecture, toutes les demandes de précision étaient renvoyées par le Gouvernement à la Conférence nationale des territoires, au cours de laquelle une concertation avec les élus locaux En réalité, l'amendement du Gouvernement était déjà rédigé pour la nouvelle lecture prévue le lendemain même à l'Assemblée nationale. Les marges de manoeuvre de la Conférence nationale des territoires étaient par conséquent très limitées, et la tenue de cette conférence s'est apparentée à une opération de communication du Premier ministre, laissant à penser que les élus gardaient tout de même la main. Il s'est agi en réalité d'un écran de fumée, conduit l'Association des maires de France à refuser d'y participer, aucun « pacte de confiance » n'étant, selon elle, aujourd'hui envisageable. Dans ces conditions, nous pouvons nous interroger sur une méthode introduire en nouvelle lecture un amendement de six pages, au contenu largement normatif, alors que les lois de programmation sont censées être indicatives ... Une nouvelle fois, avec Emmanuel Macron, nous sommes dans le marketing politique : il s'agit de vendre son produit en deux fois en faisant croire à une concertation, alors que le détail de la contractualisation, qui était déjà dans les cartons du Gouvernement, aurait pu figurer dans le texte initial, être débattu dès la première lecture, puis amendé au cours de la navette. Peut-être un compromis aurait-il même pu alors être trouvé en commission mixte paritaire, dans un esprit constructif. Les marges de manoeuvre en nouvelle lecture, avec un texte profondément remanié par des amendements gouvernementaux, sont désormais plus réduites. Il apparaît ainsi inédit incongru, pour ne pas dire abscons, que la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation ait échoué, au motif notamment que le texte serait détaillé et un compromis peut-être trouvé le lendemain, lors d'une réunion extérieure au Parlement. À l'issue de la Conférence nationale des territoires, la nouvelle mouture du projet de loi de programmation présentée par le Gouvernement reprend certaines propositions du Sénat. Cependant, beaucoup de points essentiels demeurent insatisfaisants.

Certes, cet effort sera réalisé dans le cadre d'une contractualisation proposée par l'État, mais son caractère léonin rétablit de fait une tutelle sur les collectivités territoriales. Si le contrat imposé par l'État n'est pas respecté, une reprise financière sera opérée, et si la collectivité refuse de signer le contrat, la sanction sera plus lourde encore. L'objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales retenu par le Gouvernement afin de réaliser 13 milliards d'euros d'économies sur cinq ans est donc de 1,2 % par an en valeur, comme dans le texte initial.

représente un effort, pour les collectivités territoriales, de l'ordre de 21 milliards d'euros, et non de 13 milliards d'euros. L'objectif d'une baisse de 13 milliards d'euros des dépenses des collectivités territoriales sur le fondement d'hypothèses d'évolution tendancielle de la dépense locale plus sincères avait conduit la commission des finances du Sénat à fixer l'objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à 1,9 % par an, au lieu de 1,2 %. Nous regrettons que ce taux n'ait pas été retenu. 1,2 % pourra être revu à la baisse ou à la hausse pour chaque collectivité territoriale qui contractualise, en fonction de trois critères. Si la prise en compte dans ces critères de la démographie et des efforts déjà réalisés avait été proposée par le Sénat, le Sénat, celle des nouvelles normes imposées par l'État n'a pas été retenue, ce qui était pourtant essentiel. Concernant les départements, le Gouvernement a repris la proposition du Sénat de déduire les allocations individuelles de solidarité, dont l'évolution n'est pas contrôlable par les conseils départementaux, de l'évaluation de l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Mais les dépenses liées à la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés, dont le coût est croissant, ne sont pas prises en compte, ce que nous regrettons vivement. Nous regrettons également que la sanction financière en cas de non-respect du contrat soit particulièrement lourde, avec une reprise financière de 75 %, et même de 100 % pour les collectivités territoriales concernées par la contractualisation qui auront refusé de signer Cela s'apparente à une baisse des dotations déguisée. Nous regrettons également que le dispositif du bonus soit très peu détaillé. Il est juste précisé que, en cas de respect des objectifs contractuels, le préfet pourra accorder aux communes et EPCI signataires une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l'investissement local ». Mais il s'agit d'une simple possibilité. Un contrat est pourtant censé engager les deux parties. De surcroît, le flou est total quant au pourcentage de majoration. En outre, monsieur le secrétaire d'État, des départements et des régions ? Nous nous félicitons toutefois de la prise en compte de la suppression par le Sénat de la « règle d'or renforcée à savoir le contrôle de la capacité de désendettement des collectivités territoriales : cet objectif est désormais incitatif et non plus contraignant. Cette nouvelle règle prudentielle fondée sur la capacité de désendettement faisait en effet peser le risque d'une véritable tutelle de l'État sur le recours à l'emprunt, avec des conséquences réelles sur l'investissement local. Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, ce texte qui nous revient de l'Assemblée nationale comporte encore trop d'éléments insatisfaisants. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains soutiendra et votera les amendements présentés par notre commission des finances, dont l'adoption permettra d'assurer un meilleur équilibre entre responsabilité et liberté des collectivités territoriales. La parole

du groupe Union Centriste, nous estimons qu'il s'agit plutôt d'un exercice de style, assez théorique. Comme lors du quinquennat de François Hollande, on nous promet, en début de mandat, un retour à l'équilibre en cinq ans.

L'Assemblée nationale n'a pas non plus entendu les arguments du Sénat sur l'impôt sur la fortune immobilière, qui frappera l'avertissement productif alors même que des investissements totalement improductifs seront exclus de l'assiette de l'imposition. On peut aussi regretter

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d'un calendrier parlementaire chargé.

ancrées dans le texte : c'est le cas du relèvement du taux de TVA à 10 % pour la plupart des opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement. D'autres mesures importantes ont été conservées, comme celle qui, à l'article 4, vise à préciser le régime de calcul de la TVA pour la presse en ligne. Sur ce dernier sujet, comme sur l'évolution économique en général, le Sénat montre son engagement en faveur de la nouvelle économie. Nous avons su, de manière transpartisane, mettre sur la table et discuter des mesures qui, même si elles n'ont pas toutes été adoptées, serviront de base aux textes futurs- je pense en particulier aux dispositions issues du rapport du Sénat relatif à la fiscalité de l'économie collaborative.

Nous sommes tous ici les premières cibles lorsque le Sénat s'entête dans une posture politique. Bien sûr, il n'y aura pas d'accord avec l'Assemblée nationale.

souhaite proposer aux Français l'image d'une seconde chambre qui relit, corrige et peaufine, nous voterons contre cette motion.

Je vais suspendre la séance afin de permettre à la commission des finances de se réunir pour examiner les amendements déposés sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La parole est à M. le président de la commission.

Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect des uns et des autres, ainsi que celui du temps de parole, afin que chaque orateur puisse bénéficier de la diffusion complète de sa question et de la réponse. La parole La parole est à Mme Valérie Létard, pour le groupe Union Centriste.

et au terme d'un débat budgétaire douloureux, voire décevant, sur un sujet ô combien cher à nos collectivités et à nos concitoyens, celui du logement, de son financement et de sa nécessaire réforme.

sera véritablement pris en compte et nourrira le projet de loi que le Gouvernement déposera au printemps prochain ? Pouvez-vous nous garantir que cette concertation ne sera pas qu'un prétexte pour faire accepter l'inacceptable ? Nous comptons sur vous, monsieur le Premier ministre, et sur le Gouvernement.

Vous êtes une spécialiste reconnue du sujet ;

Ces propos sont inacceptables. En luttant contre un seul ennemi, Daech, notre pays a été cohérent depuis le début du conflit syrien. Comme l'a justement précisé le Président de la République, nous ne pourrons construire de paix durable ou parvenir à une solution politique sans la Syrie et les Syriens. Mais les propos tenus par Bachar al-Assad ne semblent pas aller dans le sens de l'émergence d'une issue internationale positive pour la région. La France fait aujourd'hui partie d'une coalition internationale qui est la seule entité capable de gagner en Syrie, quand toutes les autres parties font preuve d'ambiguïtés. En conséquence, les propos de M. Assad nous paraissent tout à fait déplacés.

ennemi de son propre peuple et responsable de la mort de près de 400 000 personnes depuis le début de la guerre. Comme l'a justement affirmé le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, « quand on a passé son temps à massacrer son peuple, on a généralement un peu plus de discrétion Si nous entendons construire un processus de paix qui conduise à une véritable stabilité du pays, nous nous devons de réunir les parties autour de la table et de poser les bases d'une transition politique et démocratique durable.

bras. Il faut parvenir à embrayer sur une solution politique pour construire la paix dans la durée, comme l'a dit ce matin le Président de la République, en ajoutant que des initiatives seront prises dans le cadre du processus que la France souhaite voir émerger au début de l'année prochaine.

L'audiovisuel public fait actuellement l'objet de toutes les attentions, avec 80 millions d'euros d'économies supplémentaires demandés aux entreprises du secteur, la fuite malheureuse d'un rapport qui propose la suppression de France Ô, le basculement de France 4

cela ne doit pas faire oublier la mission éducative de l'audiovisuel public. Le manque de concertation inquiète légitimement nos concitoyens, attachés au service public, ainsi que des personnels, en métropole et dans les outre-mer, qui voient les choses se dessiner au gré des articles de presse, ne sachant où se décide précisément cette réforme. Il importe donc de définir rapidement une vision stratégique et un calendrier précis pour cette réforme que nous appelons de nos voeux. Pour alimenter votre réflexion, les entreprises du secteur vous ont remis leurs propres propositions en novembre dernier. Parmi celles de France Télévisions figure le renforcement significatif du caractère régional de France 3, de ce qui existe déjà en outre-mer grâce aux neuf chaînes du réseau Outre-Mer 1, chaînes de proximité de plein exercice. J'aimerais aller un peu plus loin et connaître la philosophie de votre ministère sur la valorisation et le partage en métropole des cultures des outre-mer pour tous les publics. Sur le fond, avez-vous retenu certaines des propositions formulées par France Télévisions, notamment en matière de régionalisation ? Nous confirmez-vous que la suppression de France Ô est définitivement écartée et que cette chaîne conservera sa vocation dans le groupe ?

de l'audiovisuel public. La présence de France Télévisions sur l'ensemble des territoires ultramarins au travers du réseau des chaînes Outre-Mer 1 est une force de notre service public audiovisuel sur laquelle nous devons nous appuyer davantage. Concernant France Ô, il est de la mission du service public de faire connaître au plus large public les actualités, la création, le patrimoine et les cultures de ces territoires. Ces dernières années, cette mission était principalement assurée par France Ô, dont la ligne éditoriale a été recentrée sur sa vocation ultramarine. En réalité, la véritable question est celle de la présence des outre-mer sur toutes les antennes nationales de France Télévisions, afin notamment de leur assurer une plus grande visibilité. Cela vaut en matière d'information comme de création audiovisuelle. Je veux d'ailleurs saluer ici la qualité des fictions et des documentaires produits par le service public sur les territoires ultramarins. Ces contenus mériteraient d'être davantage exposés sur l'ensemble des antennes nationales. Cette réflexion s'inscrit dans le cadre des travaux sur la transformation de l'audiovisuel public que le Président de la République a appelée de ses voeux et que nous avons lancée. Je rencontrerai encore l'ensemble des directeurs

Pour l'occasion, rappelant la totale solidarité que requiert cette pratique, une cordée de 330 personnes s'est déployée le long du col de l'Échelle, là même où les panneaux « France » ont étrangement été retirés pour égarer les migrants. Après avoir échappé à l'esclavage en Libye, après avoir évité la noyade en Méditerranée, hommes, femmes et enfants entreprennent par milliers la traversée des Alpes, à peine vêtus, malgré le froid, malgré la neige qu'ils découvrent pour la première fois. Jamais depuis Hannibal la traversée des Alpes n'aura été aussi périlleuse. Mais le Gouvernement français, aveuglé par les chiffres et sans considération aucune pour la souffrance humaine, ramène à la frontière, par moins 10 degrés, ces gens à peine vêtus. Comme partout sur le territoire, associations et citoyens se mobilisent pour le respect de la vie humaine, pour que l'on ne transforme pas les Alpes en cimetière. Certains ont même été condamnés pour leur humanité. Samedi, la police était d'ailleurs là pour relever les plaques d'immatriculation des encordés

Étape supplémentaire dans l'indignité, votre circulaire du 12 décembre dernier autorise désormais la police à traquer les réfugiés jusque dans les hébergements d'urgence, provoquant l'ire des ONG. Indigne et absurde, cette mesure jettera dans les rues des gens qui, pour survivre, pourraient commettre l'irréparable.

la politique de la France n'est pas indigne. Oui, nous accueillons beaucoup de celles et de ceux qui ont droit à l'asile. Ce matin encore, j'accueillais un certain nombre de réfugiés venant du Darfour et de l'Érythrée. Mais, comme l'a dit le Président de la République, autant nous devons accueillir celles et ceux qui sont victimes de la guerre ou de persécutions politiques dans leur pays, autant nous ne pouvons accueillir l'ensemble des migrants économiques.

vous le savez, toutes les associations humanitaires protestent depuis quelques jours contre la circulaire que vous avez prise le 12 décembre dernier, donnant instruction d'opérer un tri parmi les personnes accueillies dans les centres d'hébergement d'urgence, au

Il vous reste donc onze jours, monsieur le ministre, pour donner une suite positive au voeu du Président de la République. Chaque jour, depuis maintenant plusieurs semaines, un recul sans précédent

L'objectif est de les aider à accéder à leur autonomie personnelle ou sociale ou de la recouvrer. Les centres d'hébergement d'urgence, Les centres d'hébergement d'urgence, quant à eux, permettent la mise à l'abri de toute personne pour un temps très particulier. Nous le

faire ! La parole est à M. Jérôme Bignon, pour le groupe Les Indépendants-République et Territoires.

au règlement général européen sur la protection des données personnelles- le RGPD -a été adopté mercredi dernier en conseil des ministres. L'entrée en vigueur du règlement, qui réforme en profondeur notre cadre normatif de traitement des données, est fixée au 25 mai prochain.

Le RGPD constitue pourtant une véritable révolution au service d'une meilleure protection des données personnelles : il crée un « droit à l'oubli » et à la portabilité des données pour les citoyens, il oblige les entreprises à recevoir le consentement « explicite » et « positif » des utilisateurs avant le traitement de leurs données, il contraint ces mêmes entreprises à prendre en compte des exigences relatives à la protection des données personnelles dès la conception des produits. Ce règlement permet de combler en partie le retard des régulateurs européens et nationaux sur les avancées technologiques. Je souhaite saluer ici le rôle

comment la France compte-t-elle défendre au niveau européen et international le respect de ces nouvelles dispositions, notamment par les entreprises et le gouvernement américains, qui disposent d'un quasi-monopole sur l'hébergement des données numériques ?

de 1978 à un nouveau cadre juridique européen composé d'un règlement et d'une directive, laquelle devra être transposée avant le 25 mai 2018. règlement et le texte français qui le transpose instaurent de nouveaux droits pour les citoyens, en particulier- c'est très important -un droit à l'effacement des données et un droit à la portabilité des données personnelles. Le cadre juridique sécurisé ainsi dessiné permettra de renforcer la confiance des citoyens dans l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles. Pour répondre précisément à la question que vous posez, monsieur le sénateur, il faut dire que le règlement constitue un cadre très protecteur pour l'ensemble des Européens en matière de données personnelles. Il est applicable à l'ensemble des entreprises et de leurs sous-traitants, quel que soit leur lieu d'implantation, dès lors qu'ils offrent des biens et des services à des personnes résidant sur le territoire de l'Union européenne.

les pouvoirs de la CNIL sont considérablement renforcés, puisqu'elle disposera d'un pouvoir de sanction, pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial consolidé. En cas de contentieux, les juridictions nationales et/ou européennes pourront également être saisies et intervenir par rapport aux entreprises américaines. De plus, la France a souhaité être associée au « bouclier vie privée », adopté par la Commission européenne en 2016, qui permet les transferts de données des entreprises européennes vers les États-Unis. La France a a rappelé la nécessité, pour l'administration américaine, de garantir un niveau de protection équivalent au standard européen. Ainsi, c'est une nouvelle forme de souveraineté que notre pays a promu au sein de l'Union européenne en matière de données personnelles.

et vous avez supprimé l'APL accession en zone tendue. Autant dire qu'elle a quasiment disparu, puisque seulement 5 % des ménages précédemment éligibles pourront désormais y prétendre. Ma question est simple, monsieur le ministre à la veille de l'ouverture au Sénat des travaux de la conférence de consensus sur le logement, voulue par le président Larcher et par le Premier ministre, quelle est, pour le Gouvernement, la définition des termes « consensus » et « compromis »

Le 6 décembre dernier, le président Trump a annoncé sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine, qui se trouve actuellement à Tel-Aviv et compte plus de 1 000 agents.

et en instituant un rapport de force inégal en défaveur des Palestiniens. Il montre aussi le peu de cas qu'il fait de ses alliés - si l'on peut dire ! -de l'OTAN. Les Les États-Unis perdent en même temps leur statut de médiateur au Proche-Orient. Le Président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé la désapprobation de la France, en qualifiant cette initiative

La France est l'amie des Palestiniens comme des Israéliens. C'est pourquoi elle ne peut accepter ce coup de force. Comme l'a dit le Président de la République, elle cherchera à rétablir le consensus sur la ville de Jérusalem, la paix et la reconnaissance des deux États.

je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Jean-Yves Le Drian, qui se trouve précisément avec le Président de la République et le roi Abdallah de Jordanie. Le sujet que vous évoquez est naturellement au coeur de leurs entretiens.

Elle continue naturellement à parler à l'Autorité palestinienne, ainsi qu'à l'État d'Israël, puisque le Premier ministre Netanyahou était, voilà quelques jours, en France. La France est constante dans son souhait de voir advenir véritablement deux États pouvant coexister en paix

Le Premier ministre a annoncé le 15 décembre dernier à Cahors son souhait de redynamiser les centres-villes, notamment leur offre commerciale, de plus en plus moribonde. C'était une excellente nouvelle. Cependant, le même jour, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement faisait adopter un amendement au projet de loi de finances visant à diminuer de façon drastique les crédits du FISAC, le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. C'est pourtant le seul instrument de soutien budgétaire de l'État au commerce de proximité. Le Sénat avait, quelques jours plus tôt, adopté à l'unanimité tendant à abonder les crédits du FISAC de 20 millions d'euros, afin de soutenir les communes. Ce fonds a montré son efficacité, tout particulièrement dans les zones rurales, où il a contribué à la pérennisation de la dernière activité commerciale dans plus de huit communes sur dix.

et doit faire l'objet d'une action résolue de l'État. Comment expliquez-vous le décalage entre le discours de Cahors et la réalité budgétaire ? Comment pouvez-vous

Le FISAC est un instrument financier important pour le soutien au commerce, à l'artisanat et aux services de proximité en France. Depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et son décret d'application du 15 mai 2015, une nouvelle modalité de sélection des dossiers sous forme d'appel à projets a été mise en place, mettant fin à la procédure de guichet. Elle fixe des priorités thématiques et géographiques, ainsi que des critères permettant d'évaluer les projets présentés, afin de procéder à la sélection des meilleurs d'entre eux, compte tenu des moyens disponibles. La réforme du FISAC a également permis de clarifier le rôle de chaque échelon d'instruction des dossiers, dans un souci de complémentarité des moyens mobilisés. À ce jour, trois appels à projets ont été publiés. Le troisième, financé par les dotations 2018, a été diffusé en mars 2017. Ses priorités thématiques portent notamment sur la modernisation, la diversification, l'accessibilité physique et numérique des entreprises de proximité et, en milieu rural, des commerces multiservices, des derniers commerces du secteur d'activité concerné, ainsi que des stations-service. Parmi les priorités géographiques figurent les centres-villes dévitalisés connaissant un fort taux de vacance. Le plan gouvernemental « Action coeur de ville » en faveur des villes moyennes, présenté vendredi dernier, prévoit de renforcer les interventions du FISAC au bénéfice de ces collectivités.

Au total, cette réforme consolide les bénéfices du FISAC pour le commerce de proximité et corrige des déficiences que la Cour des comptes relevait dans son rapport définitif très sévère de 2014. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour le groupe Les Républicains.

décembre, bien d'autres agences du Trésor public auront baissé définitivement le rideau. C'est ce que vous appelez la réorganisation du réseau des finances publiques. L'État poursuit donc son désengagement, son abandon des territoires ruraux et périphériques. de la trésorerie de Bresles a été annoncée, les élus locaux se sont mobilisés. Ils ont alors reçu un joli courrier de la directrice départementale, dont je vais vous lire un court extrait : « Cette mesure consiste à former sur place les fonctionnaires territoriaux à l'utilisation de l'intégralité des potentialités du site. « Par Par capillarité, les fonctionnaires municipaux pourraient alors guider les usagers dans la plupart de leurs demandes, aux horaires décidés par chacune des mairies. » Aucune compensation financière n'est évoquée ! Il s'agit donc, sournoisement, d'un transfert de compétences et d'un transfert de charges qui ne disent pas leur nom. l'État fait des économies sur le dos des collectivités et de la qualité du service public ! Monsieur le secrétaire d'État, est-il cohérent d'annoncer des milliards pour revitaliser des centres-bourgs et, en même temps, de fermer des services publics dans des bourgs déjà en difficulté ?

Elle s'impose en raison de la réorganisation territoriale, avec la mise en place de nouveaux périmètres pour les intercommunalités ou la création des groupements hospitaliers de territoire, qui impliquent de travailler à une nouvelle échelle. Elle s'impose aussi parce que nous sommes dans une recherche permanente d'efficacité et de rationalisation de l'action publique. Monsieur le sénateur, vous ne devriez le sénateur, vous ne devriez pas faire comme si les mouvements de fermeture et de réorganisation de trésoreries et de points de contact de la DGFiP étaient une nouveauté. De 2008 à 2016, 400 trésoreries ont été fermées sur le territoire,

Le premier engagement, c'est la concertation. Si, dans les exemples que vous avez cités, elle a été défaillante, je suis tout à fait disposé à en discuter avec vous. Le deuxième engagement, c'est l'accès au service, notamment par l'organisation de permanences dans les maisons de services au public, dont le nombre a beaucoup progressé, et au cours des périodes de l'année qui le nécessitent.

Le Gouvernement a lancé le programme Action publique 2022, auquel j'invite toutes les sénatrices et tous les sénateurs à participer. Nous sommes prêts à expérimenter le compte financier unique, les services facturiers, tout ce qui permettra, en partenariat avec les collectivités locales, de maintenir un service de qualité sur tous les territoires de la République.

ne valent pas moins que les Français des villes ! Ce ne sont pas des citoyens de seconde zone ! Eux aussi sont des contribuables ; vous semblez l'ignorer, je le regrette profondément.

affaires étrangères. L'Europe vit des jours sombres ; l'extrême droite est de nouveau au pouvoir dans l'un de ses États membres, l'Autriche. Vendredi dernier, M. Kurz, nouveau chancelier conservateur,

dix-sept ans, une telle alliance entre la droite et l'extrême droite avait suscité une vague d'indignation. L'Europe avait alors pris des sanctions diplomatiques, on parlait de cordon sanitaire. Les conditions d'une telle riposte n'existent plus, la nécessaire unanimité des États membres la rendant impossible. Ce n'est d'ailleurs vraisemblablement pas la bonne réponse à l'expression démocratique d'un peuple. Pour autant, nous ne comprenons pas le silence assourdissant de l'Union européenne et de la France. Si la Pologne, la Hongrie, la République tchèque peuvent se réjouir de voir le groupe de Višegrad s'élargir à un nouvel allié nationaliste et populiste, la France et l'Allemagne doivent apporter une réponse politique forte pour défendre leur conception de l'Europe. conception de l'Europe. Nous ne pouvons pas accepter que le processus de fracturation de l'Union européenne se poursuive. Nous ne pouvons tolérer que les valeurs fondamentales qui ont présidé à sa création, l'attachement à l'égalité, la liberté et la justice, qui fondent la démocratie, soient remis en cause. Nous ne pouvons concevoir que, en juillet prochain, lorsque l'Autriche assurera la présidence de l'Union pour six mois, un responsable d'extrême droite ouvertement xénophobe pilote le Conseil déterminant la politique migratoire et d'asile. Nous ne pouvons imaginer que la mise en oeuvre du socle social adopté à Göteborg soit conduite par un gouvernement qui veut réserver les emplois aux seuls nationaux. Les principes fondateurs de l'Union doivent être rappelés sans concession : tous les États membres doivent garantir l'État de droit, la démocratie, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection. Or tous les éléments d'un virage autoritaire et xénophobe de l'Autriche sont réunis. La formation de ce nouveau gouvernement autrichien est un très mauvais signal au regard de l'ambition européenne du Président de la République. Quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il prendre pour défendre l'idéal européen et lutter contre la banalisation de l'extrême droite ?

Marie, Sebastian Kurz, dirigeant du parti conservateur autrichien, arrivé en tête lors des élections législatives, a constitué ces derniers jours un gouvernement de coalition avec le FPÖ, qui a été investi lundi dernier.

de maîtrise et de mise en déclin de la dette publique, l'objectif, ambitieux, étant de faire de notre pays un bon élève de la classe européenne ... Le moins que l'on puisse dire, c'est que la démarche prend un tour particulier après les deux derniers

» En effet, l'absence de compensation équitable par l'État des compétences transférées aux collectivités locales a entrainé de lourdes contraintes budgétaires, contredisant le principe d'autonomie financière des collectivités. On a apporté ici, à plusieurs reprises, la démonstration que le total de la dette de bien des départements était précisément égal

C'est pourquoi, dans le dialogue qui va se matérialiser en une proposition de contrat entre le représentant de l'État et la collectivité, il serait intéressant de faire figurer le défaut de compensation par l'État de l'exercice de ses compétences par les collectivités, ce qui permettrait de nourrir la discussion budgétaire dans les assemblées qui régissent lesdites collectivités.

un certain nombre de dispositions concernant en particulier les allocations individuelles de solidarité des départements. Le Gouvernement, dans le cadre du premier dialogue que nous avons eu à Cahors, à Cahors, a accepté de prendre en compte la spécificité des départements, qui s'étaient justement vus transférer un certain nombre de charges, en matière notamment d'allocations individuelles de solidarité. C'est donc un vrai sujet.

un total de dépenses réelles de fonctionnement de plus de 60 millions d'euros. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour le souligner, après la Conférence nationale des territoires, les modalités de contractualisation ont été précisées et très certainement améliorées,

puisse être ajusté, à hauteur de 0,15 point par critère, pour tenir compte des efforts réalisés, de l'évolution démographique et de la richesse fiscale. Nous avons fait en sorte- M. le rapporteur général vient de le rappeler

va s'engager un dialogue entre le Gouvernement et les départements, et vous évoquez une modération de la croissance des allocations. Je souhaiterais que M. le secrétaire d'État et vous-même nous disiez maintenant,

ce que représente l'apport de l'État pour l'exercice des compétences départementales, en particulier les AIS, et ce que l'on demande au contribuable départemental, c'est-à-dire le propriétaire de logement départemental.

En effet, la totalité de l'évolution des dépenses d'allocations individuelles de solidarité n'est pas prise en compte dans ce cas, ce qui posera de sérieux problèmes aux départements.

de manière à éviter de sanctionner, positivement ou négativement, un choix de gestion. En effet, selon qu'une collectivité fait le choix d'une délégation de service public ou d'une gestion en régie d'un service public à vocation industrielle ou commerciale, le niveau de ses dépenses ou de ses recettes réelles de fonctionnement

la contribution au redressement des finances publiques était calculée à hauteur d'environ 2 % des recettes réelles de fonctionnement- je parle des deux années pleines. Le risque d'une optimisation et d'une volonté de diminuer le niveau des recettes réelles de fonctionnement des budgets principaux, puisqu'il ne s'agissait là aussi que des budgets principaux, existait déjà.

de ne pas voir leurs dotations baisser, mais aussi aux 36 000 autres collectivités de France de bénéficier de la même stabilité de dotations. Il s'agit donc aussi d'un principe de confiance.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, cher Philippe Bonnecarrère, mesdames, messieurs les sénateurs, nous abordons, à l'occasion de cette session parlementaire automnale particulièrement chargée pour le ministère de l'intérieur, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Délibéré lors du conseil des ministres du 22 novembre dernier, le texte dont nous débattons aujourd'hui a pour objet de transposer deux directives et de tirer les conséquences d'une décision. tout d'abord de transposer la directive du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union Mon collègue Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, vous en présentera dans quelques instants l'économie générale. Le terme de transposition de cette directive, fixé au 9 mai 2018, commandait l'urgence de l'examen parlementaire de ce projet de loi. Il s'agit ensuite de transposer la directive du 17 mai 2017 modifiant la directive de 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Il s'agit enfin de transposer la décision du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. S'agissant de la directive du 17 mai 2017, dont le terme de transposition est fixé au 14 septembre 2018, elle a été prise sur l'initiative de la France, à la suite des attentats de Paris au mois de janvier 2015. Son fil conducteur est le renforcement du contrôle de la circulation et du commerce des armes à feu, notamment des plus dangereuses, ainsi que de la coopération intraeuropéenne sur les flux d'armes à feu. Elle a donc pour finalité le renforcement de la sécurité publique. Cette directive supprime tout d'abord la catégorie D des armes à feu, qui correspondait au régime administratif de l'enregistrement. Désormais, toutes les armes à feu devront au moins relever de la catégorie C, soumise à une déclaration, à l'exception des armes historiques et de certaines reproductions de ces dernières. La directive surclasse par ailleurs certaines armes, qui étaient jusqu'alors soumises à autorisation, pour les faire passer sous un régime d'interdiction.

et la sécurité privée, selon des modalités qui seront précisées par décret. À ce stade de mon propos, je tiens à rappeler que la directive prévoyait également la possibilité d'une troisième exception pour les collectionneurs, dans laquelle nous n'avons pas souhaité nous engager, là aussi, pour des raisons de sécurité publique. La directive impose, pour les ventes d'armes à distance, une vérification, préalable à la livraison, de l'identité et du titre de détention de l'acquéreur. En pratique, les ventes entre particuliers devront faire l'objet d'une vérification par un professionnel, préalable à la livraison, pour s'assurer de l'identité de l'acquéreur et du fait qu'il n'est pas interdit de détention de port d'armes. Enfin, le projet de loi permet aux armuriers de refuser, légalement, de conclure des transactions d'armes ou de munitions qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspectes, leur assurant ainsi une protection juridique qui fait aujourd'hui défaut. Ces dispositions sont toutes guidées par le souci de renforcer les contrôles sur la circulation et le commerce des armes, dans un but exclusif de sécurité publique. Je ne m'étendrai pas sur la nécessité et l'urgence d'insérer au plus vite de telles dispositions dans notre droit au regard du contexte que connaît notre pays, comme d'autres pays européens,

en un système de positionnement par satellites entré en service le 15 décembre 2016. Depuis lors, le lancement de nouveaux satellites se poursuit

le système Galileo émet un signal sécurisé de haute précision, le service public réglementé, dit « PRS », exclusivement réservé aux utilisateurs autorisés par décision gouvernementale. Ce signal chiffré, protégé contre le brouillage et le leurrage, est destiné à des utilisations nécessitant une grande fiabilité du signal et qui sont contrôlées par les États. À cet égard, le projet de loi nous dote des outils juridiques nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de contrôle de l'accès à ce signal sécurisé. Il prévoit notamment qu'une autorisation est obligatoire pour développer, fabriquer et exporter les récepteurs spécifiques du signal PRS ou la technologie et les logiciels associés à ce matériel. Il fixe des sanctions administratives et pénales en cas de manquement à la loi. Ces mesures permettront à la France d'assurer un haut niveau de sécurité du service public réglementé dont les applications, notamment en matière de sécurité et de défense, contribueront à assurer en toutes circonstances la protection des citoyens. Elles sont aussi le moyen de sortir de la dépendance à des systèmes de positionnement satellites étrangers, dont le contrôle échappe totalement aux pays européens.

Fidèle à sa tradition d'excellence juridique, elle a, sur la proposition de son rapporteur, procédé à un important travail de précision et d'amélioration de la rédaction de certaines dispositions, auquel le Gouvernement est favorable. Qu'il me soit cependant permis, à ce stade de mon propos, de relever une petite divergence- une différence, une discordance ? -d'appréciation sur le régime juridique des reproductions d'armes historiques, sur laquelle je reviendrai lors de

menaces et les usages. Les menaces sont nouvelles, la façon dont le numérique s'est diffusé dans l'intégralité des espaces de notre vie a évolué à une rapidité extrême. Je me réjouis donc de l'échange que nous allons

Dès 2013, le législateur français a fixé des exigences en matière de sécurité informatique aux systèmes d'informations les plus critiques pour les opérateurs d'importance vitale, les OIV, avec une liste très restrictive.

a conduit à élargir le périmètre des OIV à l'ensemble des services non seulement vitaux, mais même essentiels à la société. Cela a été tout l'objet des débats européens sur la définition des services essentiels à la société. Cette occupation répond à la multiplication d'attaques de grande ampleur, mais d'intensité moyenne,

Ces règles ont été définies à l'échelle européenne. Elles seront également applicables aux plus grands fournisseurs de services. C'est le deuxième volet de ce texte. Les fournisseurs de services numériques, du fait de l'ampleur de leurs services, parce qu'ils comptent de très nombreux clients, ont une responsabilité particulière. Si l'un de ces fournisseurs de services est défaillant

puisque nous allons traiter de trois sujets différents : la cybersécurité, les armes et le système satellitaire Galileo. Préalablement, je tiens à rassurer chacun d'entre vous sur le fait que les trois parties du texte ne posent aucune difficulté de subsidiarité. La lutte contre la cybercriminalité est bien sûr un enjeu européen, comme les questions d'armes. Quant au système satellitaire Galileo, il est par essence un programme européen.

des modalités de contrôle, ainsi qu'une obligation de déclaration des incidents à l'ANSSI. Sont concernés par la directive les opérateurs économiques dits « essentiels » et les fournisseurs de services numériques.

d'intérêt vital, ou OIV. Le champ d'application des opérateurs économiques essentiels sera plus large, en raison d'une légère surtransposition dans la définition, que je vous ai signalée, et de l'intention des services du Premier ministre, que nous avons interrogés, d'aller au-delà des sept secteurs visés par la directive en y ajoutant probablement

par voie réglementaire. Vous avez déjà tous anticipé ce que je vais maintenant vous dire : le risque est fort que ce régime soit jugé contraire à la Constitution, dans la mesure où il nous semble porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines. En effet, le législateur est tenu de définir les obligations sanctionnées, nous dit le Conseil constitutionnel, « en termes suffisamment clairs et précis » et ne peut laisser cette tâche au pouvoir réglementaire.

texte porte sur la directive relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, laquelle a connu un examen difficile devant le Parlement européen. La portée de cette directive du 17 mai 2017, qui doit être transposée avant le 14 septembre 2018, 2018, doit être relativisée. Elle est en particulier sans effet sur la lutte contre le trafic illégal, puisqu'elle ne traite en réalité que de la situation des personnes qui s'inscrivent ou s'inscriront dans le cadre légal.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

pour les opérateurs économiques d'enregistrement des transactions concernant des substances susceptibles d'être utilisées à des fins de fabrication d'explosifs, à l'exemple du TATP. Dans une logique d'augmentation du contrôle des armes à feu, la directive supprime la catégorie dite « D1 » des armes à feu et élargit la catégorie A. Le Gouvernement a fait le choix d'activer des dérogations concernant les tireurs sportifs et certaines sociétés de sécurité privée bénéficiant d'un agrément. Les ventes par correspondance d'armes restent licites, à condition que les armes soient livrées par l'intermédiaire d'un armurier ou que la plateforme utilisée soit celle d'un armurier. C'est le respect de l'obligation de déclaration qui est recherchée ; Mme la ministre vient d'en parler. Elle a également

consistant à garder les collectionneurs d'armes ou de répliques d'armes historiques dans le cadre d'un volet législatif, sans priver l'autorité publique de la possibilité d'intervenir en fonction de leur niveau de dangerosité. quelques mots concernant Galileo, le programme européen de radionavigation et de positionnement par satellites, à comparer avec le système américain GPS et les systèmes, déjà opérationnels, russes et chinois. Galileo comprend trois services distincts : un service ouvert, accessible à tous, conçu pour servir de support aux applications de géolocalisation

La décision du 25 octobre 2011, dont la transposition vous est aujourd'hui demandée, précise que, pour activer le service public réglementé de Galileo- 23 satellites à l'heure actuelle, sur 30 prévus,

Le Parlement, mes chers collègues, ne peut que donner son feu vert à la mise en oeuvre du service public réglementé. Il serait regrettable que notre défense ne puisse pas accéder à Galileo. Pour cela, un cadre minimal est

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

L'actualité récente a montré que tous les secteurs d'activité pouvaient être victimes de cyberattaques susceptibles de ralentir, voire de paralyser l'activité économique et sociétale de l'État et, bien au-delà, de compromettre la stabilité et la prospérité économiques de l'Europe.

des opérateurs de services essentiels, afin de garantir la continuité des échanges au sein du marché intérieur et la compétitivité de l'Union européenne dans le commerce international. Les cyberattaques visent aussi les fournisseurs de services numériques, lesquels jouent un rôle clef en raison de l'importance croissante du numérique. Ces services sont eux-mêmes souvent utilisés par les opérateurs de services essentiels. Il est donc primordial d'en renforcer la sécurité.

Les dispositions ainsi prévues sont parfaitement adaptées à la situation actuelle. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui assure la défense et la sécurité des systèmes d'information, a donc par nature vocation à être au coeur du dispositif de transposition. Elle se verra ainsi attribuer de nouvelles missions. J'en viens à la directive relative aux armes à feu. Elle comporte principalement des mesures visant à mieux encadrer les régimes légaux d'acquisition et de détention des armes, d'une part en durcissant les règles applicables

et le nouveau régime des reproductions des armes historiques. L'objectif du projet de loi est d'aligner les catégories d'armes nationales sur les catégories d'armes à feu prévues par la directive du 17 mai 2017. En effet, en France, les armes de chasse relèvent de deux catégories juridiques distinctes : la catégorie C, soumise à déclaration, ou la catégorie D1, soumise à enregistrement. La directive du 17 mai 2017 supprime la formalité d'enregistrement des armes de catégorie D1 pour la remplacer par la procédure de déclaration, afin de contribuer au renforcement de la sécurité publique. il n'existe plus que trois catégories d'armes à feu : A, B et C. En outre, cet alignement a pour conséquence positive de supprimer la distinction entre deux procédures administratives qui étaient, de fait, devenues semblables après les modifications introduites par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. 2016. Les chasseurs peuvent être rassurés : le changement sera administrativement neutre, plus formel que réel en quelque sorte. Quant aux armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions, elles sont actuellement classées par la loi en catégorie D2, armes dont l'acquisition et la détention sont libres.

Le projet de loi indique que les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions, seront classées par décret en Conseil d'État. En englobant toutes les armes de l'article L. 311-3, c'est-à-dire non seulement les reproductions d'armes historiques, mais également les armes historiques elles-mêmes, le projet de loi excède le champ de la directive, qui ne vise qu'à « surclasser » les reproductions d'armes historiques présentant un niveau élevé de dangerosité. Or, pour les collectionneurs, la suppression de la catégorie D mettrait les armes historiques et leurs reproductions « à la merci du pouvoir réglementaire pour reprendre leur expression. Dans ce contexte, sur l'initiative du rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement de compromis visant à conserver le classement des armes historiques et de leurs reproductions en catégorie D2, comme le demandent les collectionneurs, sauf pour certaines armes présentant une dangerosité élevée et dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État.

Il aura des applications dans une grande variété de domaines, pour des usages gouvernementaux, mais aussi dans la vie quotidienne des citoyens européens. Ce programme comprend trois services distincts : un service ouvert, accessible à tous et gratuit ; un service commercial, et un service public réglementé, le SPR, très sécurisé et à usage plus restreint.

mise en place d'une procédure d'autorisation, homologation des récepteurs, etc. Ce dernier type de contrôle incombe aux États membres, en vertu de la décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011. L'article 22 du projet de loi prévoit donc d'inscrire dans le code de la défense les dispositions de la décision du 25 octobre 2011, afin de fixer un cadre administratif minimum et préalable, ainsi qu'un régime de sanctions pénales. Dans l'ensemble, ce projet de loi se révèle conforme aux textes européens qu'il vise à transposer. Au cours de son examen en commission, aucune difficulté concernant le partage entre le domaine réglementaire et le domaine législatif n'a été constatée. Aussi le groupe Les Indépendants - République et

qu'il s'agisse de la lutte contre la cybercriminalité, du renforcement du cadre de la commercialisation des armes à feu, ou encore de l'exploitation des données collectées par Galileo. Les contraintes qui encadrent notre mission de transposition ne doivent pas nous dispenser d'un examen méticuleux des dispositions transposées dans notre droit. À cet égard, notre rapporteur a, il faut le souligner, apporté de nombreuses améliorations au texte initial. Dans ces cas précis, la transposition comporte bien des embûches. Notre rapporteur a par exemple souligné les conséquences problématiques de la suppression pure et simple de la référence des armes de catégories D proposée par le Gouvernement, ou encore la nécessité de prendre en compte les exigences constitutionnelles s'imposant aux mises en demeure préalables au prononcé d'une sanction. Nous soutenons ainsi l'essentiel des modifications qu'il a méthodiquement apportées, bien que certaines modalités de mise en oeuvre des dispositions fixées par la directive méritent quelques débats. Comme aurait pu le dire Georges Clemenceau, la cybersécurité est une chose trop grave pour la confier à des ingénieurs ! Ce sujet a été trop longtemps abandonné aux concepteurs et aux techniciens des systèmes d'information. Nous en prenons aujourd'hui progressivement la mesure, à l'occasion de piratages spectaculaires affectant nos institutions et notre économie. Aujourd'hui, le directeur de l'ANSSI nous appelle à nous saisir du problème. Selon lui, « la cybersécurité est l'affaire des décideurs Selon les estimations de la Commission européenne, l'ampleur de ces phénomènes est sans précédent : 80 % des entreprises européennes en seraient victimes, et dans certains États membres, la cybercriminalité représenterait 50 % des infractions constatées. Les victimes collatérales sont l'ensemble des utilisateurs des services affectés. Certains subissent même les inconvénients de résider dans une zone blanche tout en étant exposés à la cybercriminalité, ce qui est une situation particulièrement injuste et paradoxale, vous en conviendrez Face à l'augmentation de ces incidents, quelle réponse apporter ? La cybercriminalité aurait pu être regardée comme le prolongement électronique d'incriminations multiséculaires : le vol ou l'usurpation d'identité. Selon cette conception, le service de lutte contre la cybercriminalité aurait dû être rattaché au ministère de l'intérieur. La cybercriminalité aurait dû être combattue avec les moyens humains et matériels lui étant dévolus. En France, dès sa création en 2001, la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information a été placée sous l'autorité du Premier ministre, cette tutelle n'ayant pas été remise en cause en 2009 lors de la transformation de la direction en agence. Dès lors, l'ANSSI assure le volet préventif de la cybersécurité et le système judiciaire le volet répressif. Cette architecture institutionnelle n'est pas anodine et a influencé certaines des dispositions du projet de loi, au-delà des objectifs fixés par la directive. En premier lieu, le texte confie de nombreuses prérogatives au Premier ministre. Il nous semble qu'il aurait été plus judicieux de confier ces missions à l'ANSSI, compte tenu du nombre de décisions qui reviennent par ailleurs au chef du Gouvernement. Cela aurait permis de ne pas remettre en cause la légitimité de l'Agence en la matière, bien que, à terme, son indépendance pourrait être envisagée. En second lieu, les modalités de contrôle de l'application des normes élaborées par l'ANSSI ne sont pas satisfaisantes. Nous considérons que l'ANSSI, qui soutient déjà considérablement les opérateurs d'importance vitale, est suffisamment dimensionnée pour effectuer les contrôles nécessaires auprès des opérateurs de services essentiels publics, sans que la charge de ces contrôles incombe à ces derniers. À tout le moins, un traitement différencié aurait pu être appliqué selon la nature publique ou non des OSE, afin de ne pas mettre en difficulté des établissements publics aux finances déjà fragiles. Je pense en particulier aux hôpitaux. Enfin, en raison de la grande sensibilité des données économiques et individuelles en jeu, il nous semble que le non-respect des règles fixées par l'ANSSI devrait être strictement sanctionné, comme le prévoit la directive. Sans que les deux directives soient liées, la lutte contre la détention illégale d'armes n'est pas éloignée des questions « cyber », tant le est devenu une plateforme de fournisseurs pour les organisations de criminalité organisée. La seconde directive s'inscrit donc dans la continuité de la déclaration de Paris et des dispositions de la loi du 3 juin 2016 relatives aux armes à feu. Le régime de l'enregistrement des armes de type D1, vidé de sens, fusionne avec celui de la déclaration. La livraison d'armes est mieux encadrée, de même que la profession d'armurier, grâce aux amendements de notre rapporteur. Il serait cependant naïf de croire que ces modifications assécheront les réseaux d'approvisionnement des organisations terroristes si l'ensemble de nos partenaires européens ne s'astreint pas à une rigueur comparable.

Enfin, le surclassement des fusils à canon lisse utilisés pour la chasse pourrait placer leurs utilisateurs dans une situation d'insécurité juridique. Nous attendons donc du Gouvernement qu'il se positionne clairement sur les solutions déjà envisagées dans l'étude d'impact et qu'il donne de sérieux gages aux personnes concernées. Au-delà des réserves que je viens d'exprimer, je considère, comme la plupart des membres du groupe du RDSE, que ces transpositions constituent des avancées. Nous voterons donc ce texte. La

En matière de sécurité, l'entreprise est une cible d'autant plus exposée qu'elle est insérée dans un ensemble d'interdépendances nationales et internationales. Les menaces pesant sur les États et sur les entreprises sont protéiformes : cybercriminalité, espionnage économique, ou bien encore actions d'influence, de désinformation, de déstabilisation, atteinte à la réputation, mais aussi risques technologiques, environnementaux, sabotages. C'est pourquoi les pouvoirs publics doivent être en mesure de proposer aux entreprises françaises et européennes, ainsi qu'aux entreprises étrangères implantées en France, un niveau de sécurité suffisant pour préserver leurs intérêts et leurs richesses. Je suis fort satisfaite que la gouvernance européenne s'applique non pas uniquement dans les rapports de force entre les territoires, mais également dans un « cyber territoire dont l'aire est en réalité planétaire, et qu'elle puisse s'attacher à proposer un socle commun aux États membres. La directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, que nous transposons aujourd'hui dans notre droit, a été conçue dans cet objectif, afin d'intensifier la coopération entre les États membres sur la question essentielle de la cybersécurité. Elle établit des obligations en matière de sécurité, tant pour les opérateurs fournissant des services essentiels dans des secteurs décisifs tels que l'énergie, les transports, la santé et la finance, que pour les fournisseurs de services numériques. Veiller à la sécurité des réseaux en identifiant les risques et et créer une obligation de notification des incidents graves survenus, cela permettra indéniablement d'améliorer la sécurité de tous. Dans ce « cyber monde », lorsqu'une faiblesse est constatée sur un maillon, c'est l'ensemble des services interconnectés qui sont en réalité atteints. Il me paraît néanmoins essentiel que toutes les garanties soient apportées afin de préserver les secrets industriels et commerciaux. Sur ce point, notre rapporteur, Philippe Bonnecarrère, nous a rassurés, et j'en suis pleinement satisfaite. satisfaite. Il nous a également proposé d'apporter des précisions dans les définitions transposées, pour plus de clarté. Cela nous semble nécessaire lorsqu'on touche aux libertés publiques. La France ne part pas de rien, puisqu'elle s'est déjà dotée d'outils éprouvés et d'une agence dédiée à cet effet, l'ANSII, véritable autorité en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information pour la sécurité numérique de la nation. Cette agence nationale permet à chaque acteur d'accroître sa vigilance dans cet espace ouvert, confronté aux cybermenaces. Je formule le voeu que son rôle soit renforcé. Longtemps restée l'affaire de spécialistes, la cybersécurité est aujourd'hui un défi pour chacun d'entre nous, pour la science, pour l'industrie, donc pour l'État. l'État. Je compléterai mon propos en évoquant également un point de la seconde directive sur le contrôle de l'acquisition et de la détention des armes à feu détenues par les collectionneurs. Si le Conseil d'État nous avait rassurés dans son avis sur le cas des armes historiques et de certaines de leurs reproductions, qui demeurent en dehors du champ d'application de la directive, je salue l'initiative subtile de notre rapporteur, qui permet que ces armes soient classées en catégorie libre d'acquisition et de détention, à l'exception de certaines, dont la dangerosité serait avérée et dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État. Les collectionneurs peuvent donc être rassurés par cette mesure extrêmement protectrice de leur statut, qui leur évite des formalités fastidieuses et des restrictions sans commune mesure avec la dangerosité des armes et matériels qu'ils détiennent. La garantie de la sécurité et de l'intégrité de chaque citoyen constituant un droit fondamental, il paraît primordial que l'usage, la détention et la commercialisation d'armes à feu soient définis selon les mêmes termes dans l'espace européen de libre circulation. L'actualité nous démontre au quotidien la nécessité de raisonner au-delà de nos frontières et d'agir avec nos partenaires européens. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais adjointe au maire de Tourcoing, ville frontalière, chargée de la sécurité. Je travaillais au quotidien avec les autorités belges voisines ; c'était une nécessité locale. Je voudrais conclure en vous signalant que jeudi dernier, le général Marc Watin-Augouard, fondateur et délégué du Forum international de la cybercriminalité, nous a réunis autour des enjeux stratégiques de cybersécurité et de cyberdéfense pour préparer la prochaine édition du FIC, qui se tiendra à Lille, en janvier prochain. Vous y êtes tous invités, je pense, par la gendarmerie. J'ai donc pu à cette occasion constater à nouveau que la gendarmerie nationale était efficace et prête à s'organiser avec ses homologues européens,

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les projets de loi, présentés sous l'acronyme générique DDADUE, dont le contenu est généralement très aride, visent à incorporer à notre droit national un ensemble de directives et de règlements européens récemment adoptés. En l'occurrence, celui qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de transposer deux directives du Parlement européen et du Conseil l'une consacrée au combat pour la cybersécurité et qui doit être transposée par les États membres avant le 9 mai 2018, l'autre, destinée à lutter contre le trafic d'armes, dont le délai limite de transposition nationale est quant à lui fixé au 14 septembre 2018. Ce projet de loi tire également les conséquences d'une décision du 25 octobre 2011, relative au système de positionnement par satellites Galileo. En préambule, je voudrais souligner les progrès incontestables effectués par notre pays ces dernières années pour sortir de ce statut de « mauvais élève » en matière de transposition. À ce titre, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, ce qui démontre sa volonté d'agir vite afin de garantir un niveau de sécurité élevé des citoyens et de respecter ainsi ses engagements européens.

a pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de cybersécurité et d'établir un cadre formel de coopération entre États membres. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces dispositions, compte tenu de la menace croissante visant le patrimoine numérique des entreprises et les données personnelles des citoyens. Dans un monde de plus en plus connecté, les incidents sont devenus légion. Si la transformation numérique offre aux entreprises un formidable levier de croissance, elle induit dans le même temps une prolifération de nouveaux risques aux conséquences économiques et juridiques majeures. Selon Bruxelles, 80 % des entreprises européennes auraient connu au moins un incident de sécurité en 2016. Ce texte dote donc la France des moyens de se prémunir contre ces cyberattaques, en imposant désormais aux opérateurs et aux fournisseurs de services numériques d'identifier les risques potentiels en matière de sécurité numérique, de prendre à leur frais les décisions qui s'imposent pour les maîtriser et d'informer l'autorité nationale compétente en la matière, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Le titre II transpose, quant à lui, une directive du 17 mai 2017, prise à l'initiative de la France à la suite des attentats de Paris qui ont endeuillé notre pays en novembre 2015, et dont l'objet est de renforcer le contrôle de la circulation et du commerce des armes à feu. Le présent projet de loi permet notamment aux armuriers de refuser de conclure des transactions d'armes ou de munitions qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspectes. On peut néanmoins regretter que la directive ne traite pas de la problématique du trafic illégal, car il est un sujet majeur de préoccupation, en particulier en ce qui concerne le terrorisme. S'agissant de la question des armes historiques actives et de leurs reproductions, la commission des lois des lois du Sénat a préféré faire le choix du compromis, en revenant sur la suppression de la catégorie D. Pourtant, la directive impose aux États membres, en raison des techniques modernes qui peuvent augmenter la dangerosité des reproductions d'armes à feu anciennes, de durcir le régime qui leur est appliqué. Je réfléchis à voix haute : n'est-ce pas finalement reculer pour mieux sauter ? Le titre III porte sur la décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, qui définit les modalités d'accès au service public réglementé du système mondial de radionavigation issu du programme européen Galileo de positionnement par satellite, entré en service le 15 décembre 2016. Le projet de loi introduit un cadre réglementaire assurant sa bonne utilisation et l'assortit de sanctions pénales. Enfin, les deux derniers titres comprennent des articles non moins non moins importants, puisqu'ils permettent l'application de la loi en outre-mer et prévoient des dispositions transitoires. Ce texte a le mérite de mettre la France en conformité avec ses engagements européens. il offre à ses citoyens un espace ouvert et unifié par des législations harmonisées en matière de sécurité, dont on a malheureusement pu constater ces dernières années l'impérieuse nécessité. C'est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe La République En Marche apporteront leur entier soutien au projet de loi de transposition. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit aujourd'hui a pour objet de transposer ou de mettre en oeuvre des directives ou décisions européennes dans notre droit. Si le temps qui m'est imparti ne me permet malheureusement pas de revenir en détail sur chacune des très nombreuses dispositions de ce texte, je souhaiterais toutefois formuler quelques remarques d'ordre général. La première porte sur le déclenchement de la procédure accélérée, qui est souvent regrettable, plus particulièrement s'agissant d'un texte aussi dense et complexe. Permettez-moi, mes chers collègues, de vous citer, pour illustrer mon propos, un passage des conclusions de la commission des lois : « Tout en relevant le risque d'inconstitutionnalité de l'article 6 du du projet de loi qui, en raison de son manque de précision, pourrait être jugé contraire au principe de légalité des délits et des peines, la commission n'a pas été en mesure d'y apporter des améliorations, les consultations portant sur le socle minimal de mesures de sécurité à imposer aux opérateurs économiques essentiels n'étant pas achevées au niveau interministériel ». Édifiant, n'est-ce pas ? Par manque de temps pour travailler de manière satisfaisante, la commission se contente de « relever » le risque d'inconstitutionnalité. Ensuite, quel besoin y avait-il de traiter de trois sujets distincts, mais d'égale importance dans un même texte ? La cybersécurité, la réglementation sur les armes à feu civiles et le système de positionnement par satellite Galileo recouvrent des enjeux bien différents qui auraient mérité d'être traités séparément dans un temps propice à un travail parlementaire de meilleure qualité. Faut-il le rappeler, mes chers collègues, nos concitoyens font preuve d'un véritable désamour à l'égard de l'Europe et de ses institutions, qu'ils envisagent au mieux comme une bureaucratie intrusive, au pire comme un instrument supplémentaire de paupérisation. Plutôt que de faire preuve de pédagogie, de montrer la nécessité de construire, ensemble, un socle de droits et de devoirs cohérents, nous examinons, pardonnez ma familiarité, à la va-vite un texte quelque peu fourre-tout. Sur le fond pourtant, il y avait matière à montrer que l'Europe peut être protectrice et parfois même faire fi des pressions des lobbies. Prenons l'exemple de la directive relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Ce texte, demandé par la France après les attentats de 2015, a pour objet de réduire les sources potentielles de trafic illégal d'armes à feu et de limiter l'accès aux armes les plus dangereuses. Il vise notamment à lutter contre le détournement à des fins criminelles d'armes prétendument neutralisées. ce texte existe, malgré l'intense lobbying des « proarmes » au Parlement européen, souvent relayé par les députés conservateurs et d'extrême droite, voire par certains libéraux. Comme l'a rappelé notre collègue eurodéputé Pascal Durand, dont je partage l'analyse : « Les progrès réglementaires sont le fruit d'un compromis entre les objectifs de sécurité publique, en luttant notamment contre contre les risques de trafic d'armes, et la possibilité d'acquérir une arme sur le marché intérieur. Ceci implique, entre autres, le contrôle de l'identité des personnes acquérant une arme en ligne et, de la part des États membres, le partage des informations sur la possession d'armes à feu sur leur territoire. Par ailleurs, la vérification périodique ou continue de l'aptitude psychologique à détenir une arme à feu est désormais obligatoire et des restrictions s'appliquent sur l'entreposage des armes. » Ce sont là de véritables avancées pour la sécurité commune comme pour la sécurité de chacune et de chacun, et nous nous en réjouissons. Ainsi, c'est avec le sentiment d'un travail certes pas tout à fait accompli, mais convaincu de la nécessité de poursuivre la construction d'un droit européen cohérent, que le groupe CRCE soutiendra ce texte. La parole

Face à l'inflation des cyberattaques, vous avez été nombreux à les citer, il importe de répondre rapidement et de s'adapter le mieux possible.

d'objets seront connectés dans l'UE. Dans ce contexte, le projet de loi, comme l'a souligné notre rapporteur, donne un cadre législatif à la stratégie européenne en matière de cybersécurité qui émerge progressivement et invite de fait les États à une stratégie nationale de sécurité. Dans cette double stratégie européenne et nationale- les deux niveaux sont intrinsèquement liés

pour laquelle près de la moitié des États membres ont mis en place un dispositif. Il est à noter que la France fait partie des quelques pays ayant une vraie expertise en la matière. Ce projet

de sanctions pénales. La notion de confidentialité appellera les acteurs économiques à une stratégie de certification renforcée. C'est là qu'il conviendra d'être particulièrement vigilant, sous

De la cybersécurité aux régimes des armes à feu, des armes à feu aux satellites du système Galileo, le champ que nous balayons ce soir est vaste. Je ne m'étendrai pas sur Galileo, mais je salue tout de même l'ambition de ce projet, qui permettra à terme de mettre fin à toute dépendance de l'Europe aux États-Unis en matière de positionnement par satellite. La suite de mon propos sera brève et concentrée sur les titres I et II du projet de loi. Le titre Itranspose la directive NIS du 16 juillet 2016. Rappelons que cette directive s'inscrit dans le cadre d'une stratégie européenne en matière de cybersécurité et qu'elle constitue la première initiative législative européenne ainsi que la première tentative d'harmonisation des normes dans ce domaine- il n'était pas trop tôt. Le renforcement du niveau de cybersécurité des États membres pour les activités économiques stratégiques est un enjeu majeur, vous l'avez tous largement souligné. L'accélération des progrès technologiques, notamment en matière d'objets connectés, qui nous accompagnent dans pratiquement tous les aspects de notre vie quotidienne, nous oblige à nous mobiliser à une échelle qui ne peut plus être seulement nationale. Les dégâts causés par les cyberattaques ne cessent de s'accroître. M. Philippe Bonnecarrère évoque dans son rapport le cas de l'attaque informatique subie par l'entreprise française Saint-Gobain au mois d'août 2017, qui aurait entraîné des pertes s'élevant à environ 250 millions d'euros. À la fin du mois de novembre dernier, la révélation de l'attaque dont a été victime la société Uber inquiète également : quelque 57 millions de comptes utilisateurs de la plateforme ont été piratés, dont les données de 600 000 chauffeurs de l'entreprise. Alors que cette attaque remonte à la fin de l'année 2016, l'entreprise n'avait jusqu'à présent rien dit, et avait même payé une rançon aux hackers pour que ces derniers ne révèlent pas cette énorme fuite de données personnelles ... On pourrait multiplier les exemples, et vous l'avez fait, Ce phénomène ne concerne pas uniquement de grandes multinationales. Les attaques informatiques, de plus ou moins grande ampleur, concernent aussi des entreprises de taille parfois bien plus modestes et se répercutent sur un grand nombre de citoyens. Aujourd'hui croissante au niveau de l'ensemble des trafics et parfois des plus sordides, la cybercriminalité dispose d'un champ d'action quasi illimité. La puissance publique doit réagir, s'adapter, et c'est l'objet de la directive européenne du 6 juillet 2016. Il s'agit de protéger les opérateurs de services essentiels dans les secteurs publics et privés concernant la santé, le transport, l'énergie, l'alimentation, la logistique et le social. Peut-être d'autres domaines seront-ils ajoutés. Désignés par le Premier ministre, ces acteurs essentiels au bon fonctionnement de l'économie et de la vie quotidienne appliqueront des règles de cybersécurité particulières, suivies et évolutives. Le cas Uber, que je viens d'évoquer, est un bon exemple de ce qui peut se passer quand un acteur économique est confronté à ce type d'attaque : il se tait. Il se tait de peur que sa réputation n'en soit gravement ternie, exposant par là même des milliers de citoyens empêchant aussi par son silence la réaction des services de l'État, qui est seul en situation à la fois d'enquêter sur les raisons de l'attaque, d'apporter des solutions d'urgence et, surtout, d'éviter que d'autres acteurs ne subissent le même sort. Pour ces raisons, les dispositions du présent texte imposent des règles obligeant le signalement des incidents de sécurité. Celles-ci sont fondamentales pour que l'ANSSI puisse pleinement jouer son rôle, aussi bien de manière préventive qu'en temps de gestion de crise et, bien sûr, en termes d'évaluation et d'évolution du système.

Quel est l'enjeu ? Est-ce le régime juridique applicable aux 220 000 tireurs sportifs que compte notre pays ? Ou bien les obligations à la charge des collectionneurs ? Probablement pas. Selon nous, le sujet qui doit concentrer toute notre énergie est la lutte contre le trafic d'armes. Or force est de constater que peu des dispositions qui nous sont soumises ce soir sont de nature à radicalement endiguer ce trafic, lequel alimente aussi bien la grande criminalité organisée que le terrorisme. C'est pourtant la France, après les terribles attentats qu'elle a subis en 2015, qui avait été à l'origine de la directive que nous transposons aujourd'hui. Nous sommes naturellement favorables aux dispositions prévues par le présent projet de loi, qui visent néanmoins à sécuriser les conditions de ventes d'armes à feu. dirai un mot tout de même du durcissement du régime des armes historiques. Nous avons été plusieurs à être interpellés dans nos départements sur cette question. De nombreux collectionneurs d'armes anciennes ont émis des craintes sur l'article 16 du texte, qui précise que le classement de ces armes et leurs reproductions ne relèvent plus de la loi, mais sera défini par décret en Conseil d'État. Or les armes historiques elles-mêmes demeurent en dehors du champ d'application de la directive. La commission des lois, qui a excellemment travaillé, a fort opportunément considéré que les armes historiques et leurs reproductions seront classées en catégorie D2, exception faite de certaines armes dangereuses qui seront énumérées par décret. Je tiens à remercier chaleureusement notre collègue Philippe Bonnecarrère et à le féliciter pour la grande qualité de son rapport. Moi aussi ! Il a su faire preuve de pédagogie dans la présentation de son analyse sur des sujets très techniques, notamment sur l'aspect de cybersécurité.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste, comme les autres groupes, du reste, votera en faveur du projet de loi, dans la rédaction issue des travaux de notre commission des lois. La discussion

Monsieur le ministre

51 % des citoyens européens ne se sentent pas suffisamment informés sur les risques liés aux cyberattaques et deux tiers des entreprises n'ont jamais évalué les risques financiers liés à ces attaques, selon une estimation de la Commission européenne. La directive souligne pourtant que les informations relatives aux incidents s'avèrent de plus en plus précieuses pour le grand public et pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Bien que ces incidents soient de plus en plus médiatisés, la plupart d'entre eux se règlent dans la confidentialité, avec le concours de l'ANSSI et des centres d'alerte et de réaction aux attaques informatiques déjà mis en place. La directive vise justement à renforcer la coopération de l'ensemble de ces acteurs au sein de l'Union européenne. À cette fin, elle prévoit que les OSE notifient les incidents à l'autorité compétente « sans retard injustifié une formule peu courante en droit français. Le rapporteur lui a donc préféré l'expression « sans délai après en avoir pris connaissance ». Nous considérons qu'il serait préférable de mentionner simplement que ces notifications ont lieu sans délai, ce qui serait plus conforme à l'esprit de la directive, qui vise à contraindre les opérateurs de services essentiels à adapter leurs pratiques au risque accru de cyberattaques. cyberattaques. Il est évident que la sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article 9 ne vise pas les dirigeants d'opérateurs aptes à prouver que l'incident significatif en cause était difficilement détectable. ailleurs, pour des raisons commerciales ou stratégiques, certains opérateurs pourraient être tentés de sous-communiquer ces incidents à l'ANSSI afin de ne pas perdre d'utilisateurs si cette attaque était rendue publique. C'est pourquoi nous préférons la formule « sans délai », qui ne laisse place à aucune ambiguïté. La sécurité des utilisateurs et de leurs données doit primer sur toute autre chose. Une bonne coopération serait en outre favorable à l'ensemble de l'écosystème.

pourra dans certains cas en prendre connaissance que plusieurs mois après. Voilà pourquoi nous avons retenu cette formulation. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Les deux premiers alinéas de l'article 14 de la directive contraignent les États membres à veiller à ce que les OSE, les opérateurs de services essentiels, prennent effectivement les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour la gestion des risques « cyber » et pour prévenir les incidents. Il ne s'agit pas d'une faculté pour les États membres, mais bien d'une obligation, qui, pour être effective, nécessiterait la mise en place d'un contrôle systématique des OSE, ce que ne prévoit pas la rédaction actuelle. L'amendement vise donc à adapter le texte aux exigences fixées par la directive. Sans contrôle, le respect des nouvelles exigences de cybersécurité est voué à rester théorique. Nous avons conscience que la systématisation de tels contrôles et l'application effective de ces nouvelles exigences de sécurité pourraient constituer une importante charge financière supplémentaire pour les opérateurs concernés, qui ne sont pas encore en conformité au regard de ces règles. C'est le cas notamment des établissements publics, tels que les hôpitaux, qui sont des cibles privilégiées des cyberpirates, récemment le piratage du NHS au Royaume-Uni. Sans parler des graves dysfonctionnements et des pertes humaines qu'une telle attaque pourrait occasionner, les hôpitaux accumulent également de nombreuses données personnelles qui pourraient être exploitées à des fins de rançon. C'est pourquoi nous aurions souhaité, dans le même temps, prévoir que la mise en oeuvre du renforcement de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux des établissements publics concernés soit prise en charge par l'État, de même que les contrôles conduits. Nos amendements ont malheureusement été déclarés irrecevables financièrement. Il s'agit toutefois d'une question dont le Gouvernement devra rapidement se préoccuper, de même que de l'articulation de ce dispositif avec la protection des données personnelles, particulièrement exposées aux cyberattaques. Il est d'ailleurs regrettable que les dispositions mentionnées au 4° de l'article 15 de la directive ne figurent pas dans le texte de transposition : elles prévoyaient d'associer la CNIL au traitement d'attaques touchant des données personnelles.

voix l'article 8. La parole est à M. le secrétaire d'État. L'article 11 vise à transposer l'article 18 de la directive, qui prévoit que les fournisseurs de service numérique établis hors de l'Union devront désigner un représentant dans l'un des États membres et se conformer aux dispositions prises par ce dernier pour la transposition de la directive.

un classement législatif des armes historiques et de leur reproduction. Nous émettons une première réserve sur ce point. La deuxième réserve tient au fait que la directive que nous transposons érige en principe le classement dans une catégorie contrôlée par l'État des reproductions d'armes historiques. Vous inversez la logique de la directive en posant comme principe l'absence de contrôle de l'État et en renvoyant au décret le soin de préciser d'éventuelles dérogations. Troisièmement, vous parlez de « dangerosité avérée

L'honorabilité n'impose pas de précision et de qualification législative pour qu'elle soit utilement contrôlée. Mais, si c'est pour faire plaisir à Mme Carrère, le Gouvernement